La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires

sur ce texte. Mes chers collègues, je vous rappelle que ce scrutin s'effectuera depuis les terminaux de vote. Je vous invite donc à vous assurer que vous disposez bien de votre carte de vote à vérifier que celle-ci fonctionne correctement en l'insérant dans votre terminal de vote. En cas de difficulté, vous pouvez demander

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France a attendu que les effets du réchauffement climatique se fassent ressentir avec plus de force et, surtout, que la sécurité d'approvisionnement en énergie se fragilise pour relancer enfin le nucléaire et les énergies renouvelables. Que de temps perdu ! Cela nous impose désormais de légiférer dans l'urgence pour nous mettre au pas et rattraper plus de vingt ans d'inertie afin de préserver notre souveraineté électrique.

Mais les revirements ne constituent pas une spécificité nationale : l'Allemagne et la Belgique ont repoussé la sortie du nucléaire, la Suède et les Pays-Bas procèdent à sa relance, quand d'autres pays, comme la Pologne, se lancent dans la construction de réacteurs. Mes chers collèges, le mix énergétique doit être diversifié. Je regrette que le Sénat ait remplacé cet objectif par celui de décarbonation. Les études prospectives réalisées ces dernières années le démontrent : plus la diversification est poussée, plus on maîtrise les incertitudes dans l'accès aux matières critiques, les technologies ou les coûts. Toutes les énergies décarbonées ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est un pari que nous faisons, car l'équation est complexe. Atteindre un mix 100 % renouvelable d'ici à 2050 ne serait pas réaliste. Ce serait non seulement coûteux, mais irréalisable, puisque nous ne disposons pas des moyens de stockage d'électricité nécessaires pour pallier les intermittences- même si les investissements dans l'hydrogène connaissent un coup d'accélérateur en raison du nouveau contexte géopolitique. Il nous faut préserver une certaine souplesse pour adapter nos objectifs de politique énergétique à ce contexte, aux freins sociaux, économiques et financiers, ainsi qu'au rythme des avancées en matière d'innovation, qui ne peuvent se décréter. Les choix du passé s'imposent pour l'avenir. On ne peut faire table rase d'une réalité qui, elle aussi, s'impose à nous : le mix électrique français repose à 70 % sur l'énergie nucléaire. Par ailleurs, les efforts de sobriété doivent également être poursuivis en parallèle si nous ne voulons pas sombrer dans la décroissance. En effet, les premiers réacteurs EPR 2 ne seront pas disponibles avant 2035, voire 2037, au mieux. Pour revenir au coeur du débat, ce projet de loi contribuera à accélérer la procédure administrative en matière de construction de nouveaux réacteurs et à prévenir les contentieux en limitant les occasions de former des recours dilatoires, sans pour autant modifier les règles de fond des autorisations environnementales et des autorisations de création. Le choix d'implanter des projets sur les sites existants, ou à leur proximité immédiate, renforcera leur acceptabilité, mais aussi leur réussite, les territoires étant déjà prédisposés pour les accueillir. C'est le cas de la centrale du Blayais, chère à notre collègue Nathalie Delattre. À l'issue de nos travaux, le texte a été complété, notamment par l'intégration de petits réacteurs modulaires, l'extension de la durée d'application des mesures de quinze à vingt-sept ans et la prise en compte des observations des collectivités. Les améliorations portées à la consultation du public sont bienvenues.

Enfin, si nous saluons une meilleure prise en compte du dérèglement climatique et des cyberattaques, nous regrettons que le périmètre des plans particuliers d'intervention n'ait pas été élargi, comme le proposait notre collègue Véronique Guillotin. Restons lucides : ce projet de loi ne règle en rien les retards accumulés par notre pays, qui n'a plus construit un seul réacteur depuis vingt ans. Les déboires du chantier de Flamanville doivent servir d'épouvantail. Ce texte demeure symbolique dans son contenu. Des obstacles, qui ne relèvent pas des procédures, persisteront. Outre les difficultés de recrutement à résoudre, il faudra préciser rapidement le volet relatif au montage financier. Par ailleurs, quelle régulation du marché de l'électricité sera appliquée Le mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), qui doit prendre fin en 2025, ne protège ni les consommateurs français ni EDF, lourdement endettée à la veille de sa nationalisation. Le marché de l'énergie doit être réformé. On ne peut continuer à subventionner les fournisseurs alternatifs et à favoriser la concurrence pour la concurrence, sans aucune incitation à l'investissement. Oui à la souveraineté, mais oui aussi à la solidarité au niveau européen et à plus d'équité ! En ce qui concerne le calendrier, la concertation publique arrive soit trop tôt, soit trop tard : trop tard, car elle aurait dû avoir lieu il y a quelques années ; trop tôt, car nous ne disposons pas des études de faisabilité et de la liste des sites d'implantation non plus que du coût total du programme de relance du nucléaire et de ses modalités de financement. S'il est facile d'acter des objectifs dans la loi, ceux-ci doivent être réalistes. Le débat public se poursuit actuellement et la représentation nationale aura l'occasion de s'en saisir. Que l'on y soit favorable ou non, les amendements du rapporteur visant à supprimer le plafonnement de la part du nucléaire à 50 % en 2035 ont quelque peu préempté ce débat. Cela étant, cet ajout ne constitue pas une ligne rouge pour notre groupe. Gageons que l'architecture générale des choix énergétiques de la France disposera de ses murs porteurs d'ici à la fin de cette année. Ainsi, le groupe RDSE votera en faveur du projet de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

déclare dans la presse que le Sénat n'est pas dans son rôle, qu'il préempte la discussion nationale sur la stratégie nucléaire : elle aurait souhaité que nous nous taisions

Le 10 février 2022, le Président de la République nous présente un programme complet, avec cet art oratoire si particulier qui consiste à parler interminablement sur des sujets qu'il est censé connaître parfaitement. Or cela n'est pas vrai, cela n'est pas vrai, parce qu'il aurait dû poser la question principale en matière d'énergie à ce jour : s'agit-il de décarboner ou bien de verdir ? S'il s'agit de verdir, la majorité sénatoriale considère que ce n'est plus la priorité. L'urgence climatique exige de décarboner notre société grâce aux mesures prises dans les

La parole est à M. Pierre Médevielle, pour le groupe Les Indépendants-République et Territoires. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en 1963, le général de Gaulle qualifiait déjà l'énergie atomique comme « le fond de l'activité de demain Que de chemin parcouru depuis le prix Nobel attribué à Pierre et Marie Curie, associés à Henri Becquerel, pour la découverte de la radioactivité naturelle ! Le nucléaire, c'est l'histoire de la France, de ses physiciens visionnaires et innovants. C'est une aventure industrielle, une aventure d'excellence et d'indépendance énergétique. Énergie respectueuse du climat, le nucléaire fournit en outre de l'électricité de façon continue et est capable de s'adapter aux variations de la demande électrique. de la stabilité de son réseau et de son caractère pilotable, il contribue largement à sécuriser l'acheminement de l'électricité à destination des hôpitaux, des entreprises et de chaque foyer. De notre force historique, il ne reste- hélas ! -que l'absolue nécessité de reconstruire une filière largement malmenée ces dernières années. Entre hésitations coupables et accidents spectaculaires, nous avons considérablement revu à la baisse nos ambitions dans ce secteur. Si Ségolène Royal et ses « acolytes » ont manqué de réalisme et de vision, si, collectivement, nous n'avons pas suffisamment soutenu cette filière, l'heure doit être aux choix politiques clairs et forts. N'oublions pas que nos centrales nucléaires sont la principale source d'électricité décarbonée. Malgré nos 87 % d'électricité d'origine nucléaire en 2010, nous nous sommes reposés sur nos lauriers en négligeant coupablement les autres modes de production. Nous discutons abondamment de bouquet, de mix, mais les leçons des deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979 n'ont pas été retenues et nous sommes toujours dépendants- à 70 % -des énergies fossiles. Le déclenchement de la guerre en Ukraine nous l'a cruellement

À cette occasion, nous avons entendu la principale critique derrière laquelle un certain nombre de parlementaires de tous bords se sont abrités pour ne pas voter ce texte, notamment à l'Assemblée nationale. Leur argument est purement chronologique : ils auraient préféré que la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie ait été discutée en amont. Nous sommes tous d'accord, mais l'invasion de l'Ukraine nous a conduits à une situation d'urgence énergétique absolue, qui a exigé des réponses efficaces et rapides. loi dits « d'accélération » ne sont peut-être pas complètement suffisants, mais ils sont essentiels pour redéfinir un cap pertinent. En ce qui concerne le nucléaire, ce texte, en l'état, comporte des avancées notoires en matière de simplification des procédures et de réduction des délais. Gagner du temps, ou en perdre moins, voilà l'enjeu ! Tout d'abord, nous sommes très nombreux, sur les travées de cet hémicycle, à nous réjouir de la suppression, au sein du code de l'énergie,

En outre, la recherche et l'innovation dans le domaine de l'hydrogène bas-carbone font partie de nos objectifs à long terme. Enfin, plusieurs garanties sont ajoutées concernant la sûreté et la sécurité des installations face aux aléas du dérèglement climatique. Être toujours plus transparents et prévoyants doit rester notre préoccupation essentielle. Si l'opinion publique a très favorablement évolué dans ce domaine, la pleine acceptation des Français n'est pas au rendez-vous c'est la raison pour laquelle la sécurité et la sûreté nucléaire doivent rester, plus que jamais, notre priorité. En matière de prévention, la France a placé la barre beaucoup plus haut que les autres pays. Grâce aux nouvelles évolutions technologiques, comme les réacteurs moyen-module ou le projet (Iter) ayant trait à la fusion, toutes les conditions sont réunies pour donner un véritable second souffle à cette filière qui, associée à l'énergie solaire, doit nous permettre d'atteindre, dans quelques dizaines d'années, ce graal qu'est l'indépendance énergétique.

Le manque flagrant d'équipes compétentes dans le domaine de la maintenance a considérablement ralenti la remise en service de nombreux réacteurs depuis le début de la crise énergétique. le meilleur de l'innovation reste encore à inventer et les récents succès des Américains dans le domaine de la fusion nous autorisent tous les espoirs. Enfin, le redressement de notre économie et de nos comptes publics sera directement lié à nos ambitions en matière d'indépendance énergétique. Le nucléaire est l'une des sources d'électricité décarbonée peu coûteuse à produire, permettant à la France d'avoir un prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe. N'écoutons pas les « Khmers verts » et les « prédicateurs de la lampe à huile », dont le discours irréaliste ne peut que nous conduire dans des impasses mortifères pour les générations futures. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires sera sans ambiguïté et votera ce texte, symbole fort d'un cap à tracer et à poursuivre. Excellent La parole est à M. Daniel Salmon, pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte a changé de nature. Il traduit maintenant le programme politique des Républicains, avec le consentement du Gouvernement. Un programme qu'ils auraient dû lancer lorsqu'ils étaient au pouvoir pour disposer de nouveaux réacteurs opérationnels aujourd'hui ! Si tant est que l'EPR démarre un jour ... « Ce projet de loi n'est pas une loi de programmation », avez-vous insisté madame la ministre, tout au long du parcours de ce texte au Sénat. Il n'était pas censé préempter les décisions qui seraient prises sur l'avenir du mix énergétique français. Pourtant, au détour d'un amendement, dont l'objet très vague tendait à la diversification du mix électrique en visant un meilleur équilibre entre le nucléaire et les vous avez acté,, le renoncement à l'objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Nous regrettons profondément ce recul conséquent et grave pour l'avenir énergétique de notre pays. Le nucléaire demande une stabilité à toute épreuve, alors que le monde vit, et vivra, des décennies de grandes turbulences, climatiques et géopolitiques. Ce choix dogmatique nous engage de manière irréversible pour le siècle à venir, au mépris du processus démocratique et des concertations en cours,

se désolent également de ce procédé complètement antidémocratique, qui revient à « considérer comme sans intérêt [ ...] les interrogations, les remarques et les propositions faites » par nos concitoyens.

le code de l'énergie. Nous passons ainsi du principe d'un plafond à celui d'un plancher, ce qui change tout ! Ce changement de paradigme nous engage dans un avenir particulièrement incertain. Cette mesure s'accompagne d'une palette de dispositifs en faveur d'une relance maximaliste du nucléaire, sans la moindre nuance : suppression du plafond de 63,2 gigawatts de capacité nucléaire installée ; révision du décret prévoyant la fermeture de douze réacteurs, en plus de celui prolongation de la durée d'application du texte, initialement prévue jusqu'à 2038, jusqu'à 2050 ; qualification de projets d'intérêt général, par un décret en Conseil d'État, des projets d'installations d'entreposage de combustibles nucléaires ; ou encore, durcissement des peines sanctionnant les intrusions au sein de centrales nucléaires. Plutôt que de renforcer la sécurité des centrales, on préfère s'en prendre aux lanceurs d'alerte ! Les militants de Greenpeace, à travers ces actions, dénoncent justement les problèmes de sécurité des sites nucléaires. Casser le thermomètre n'a jamais fait tomber la fièvre du malade ! En résumé, des mesures situées strictement à l'opposé de nos recommandations. Rappelons les objectifs de ce texte

ce ne sont pas les procédures environnementales qui ont fait prendre du retard à la filière. Le problème du nucléaire est bien plus profond et relève notamment d'un problème de compétences, mis en évidence par le fiasco de l'EPR de Flamanville. Clairement, nous ne cernons toujours pas l'intérêt de ce texte face à l'urgence climatique. En effet, avec de premiers réacteurs opérationnels en 2040, il sera déjà bien trop tard ! Prendre des mesures pour gagner quelques mois ne sert absolument à rien. (GIEC) ne cesse de marteler que les principaux investissements dans la transition énergétique doivent être réalisés dans les dix ans. Pourquoi n'entendez-vous toujours pas cet argument rationnel et scientifique ? Nous avançons à l'aveugle s'agissant de ce choix de construire plusieurs EPR, qui représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements. Cet argent, nous en avons besoin, maintenant, pour développer les installations d'énergies renouvelables et pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique,

Les énergies renouvelables deviennent très compétitives, et cela en incluant le coût des capacités de flexibilité et de stockage. Chaque année, elles deviennent moins chères. quant à lui, de plus en plus coûteux, sans parler des dettes laissées aux générations futures, en termes de déchets et de démantèlement. L'avenir n'est pas dans les paris technologiques qui risquent de mettre gravement à mal notre économie. Si quelques apports positifs sont adoptés, ils demeurent très à la marge. Nous notons, tout de même, à l'article 9 , l'ajout du rapporteur en faveur d'une meilleure intégration de la cybersécurité dans la sécurité nucléaire et d'une meilleure prise en compte de la résilience des réacteurs au changement climatique, lors de la demande d'autorisation de création et du réexamen décennal. Cependant, le risque de l'étude de vulnérabilité ainsi prévue est qu'elle ne porte que sur un temps très court et ne prend pas en compte l'échelle de vie du réacteur. (ASN), elle-même, estime que le pas décennal n'est pas adapté à l'anticipation des effets du réchauffement climatique. Il faut se projeter jusqu'à la fin du siècle. Seul réel motif de satisfaction : l'unique amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires adopté, tendant à renforcer notre sécurité collective, en empêchant la construction de nouvelles centrales nucléaires sur des zones littorales vulnérables aux inondations. Cette mesure de bon sens doit être absolument maintenue ! La problématique de l'eau a des effets aussi bien sur les anciennes centrales que sur le nouveau nucléaire. Le risque d'inondation ou de submersion marine comme la baisse d'étiage des fleuves dans les années à venir, largement démontrés par plusieurs rapports, sont des sujets centraux pour la sûreté et pour la protection des milieux naturels.

la modification de notre mix énergétique, et donc de notre PPE, s'ajoute au détricotage du code de l'urbanisme et du droit de l'environnement, pour de nouveaux réacteurs dont le Parlement n'a pas même encore validé le principe. Nous sommes clairement en Absurdie et sommes atterrés par tant de dogmatisme et d'aveuglement. et Territoires votera contre ce texte, qui reléguera encore davantage au second plan l'indispensable déploiement des énergies renouvelables et les investissements dans la rénovation thermique, seuls capables de répondre aux enjeux climatiques et de souveraineté. La parole est à M. Bernard Buis, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

Certains collègues ont considéré que ces débats n'étaient pas assez nourris. Pourtant, ces échanges ont surtout révélé une certaine convergence de vues entre nous sur ce texte, première pierre d'un immense chantier pour la relance du nucléaire en France. ce projet de loi de simplification des procédures est technique- très technique -ce qui a limité l'inflation d'amendements et ce qui devait,, éviter de longs débats de fond

Quelques désaccords sur le fond, qui risquent d'amoindrir la portée des articles, et une véritable divergence s'agissant de l'angle programmatique ajouté. que la majorité sénatoriale supprime l'objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici à 2035, tout en imposant la révision du décret prévoyant la fermeture de douze réacteurs. C'est sans trembler que la majorité sénatoriale supprime le plafond autorisé d'électricité nucléaire, fixé à 63,2 gigawatts, dans le code de l'énergie. Mes chers collègues, la question n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre la relance du nucléaire. À titre personnel, j'y suis très favorable. Au fond, il me semble qu'il s'agit plutôt de comprendre pourquoi vouloir balayer d'un revers de main les consultations en cours. Peut-être par impatience, afin de marquer un positionnement assumé, profitant ainsi de ce véhicule législatif pour envoyer un signal fort. Reconnaissons que, soucieux d'écouter la majorité sénatoriale, sénatoriale, le Gouvernement a fait un geste en défendant un amendement visant à un meilleur équilibre entre le nucléaire et les énergies renouvelables ; un amendement d'appel qui ne précise en rien le rapport de cet équilibre. fois encore, ce projet de loi n'est pas un texte programmatique ; l'équilibre de ce mix énergétique n'est pas- et ne sera pas -l'objet de ce texte d'accélération des procédures. Deux consultations publiques sont en cours.

Cette concertation s'est poursuivie sous la forme d'un forum des jeunesses à Paris, réunissant 200 jeunes, âgés de 18 à 35 ans, sélectionnés par tirage au sort L'autre consultation, animée par la Commission nationale du débat public, doit débattre de l'avenir du nucléaire de demain. Elle a débuté le 27 octobre et doit se poursuivre jusqu'au 27 février prochain.

D'ailleurs, sur ce point, la CNDP a été très claire, en considérant que cette anticipation de la programmation pluriannuelle de l'énergie revenait « à considérer comme sans intérêt les interrogations, les remarques et les propositions faites lors du débat public en cours pour définir la stratégie énergétique Nous attendons de la navette parlementaire qu'elle revienne sur ces dispositions, afin de respecter ce temps démocratique nécessaire à l'acceptation de notre nouvelle stratégie énergétique. Aussi regrettons-nous que le Sénat ait mis un peu de plomb dans l'aile aux objectifs de simplification du texte. Je pense, par exemple, à l'article 3 concernant la dispense d'autorisation d'urbanisme. Les précisions apportées au décret en Conseil d'État créent désormais quasiment un nouveau régime d'autorisation contre-productif. Je pense à l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cadre de la délivrance de l'autorisation environnementale, dont l'apport semble peu pertinent pour les aspects préparatoires au chantier.

dans la vallée du Rhône. À ce sujet, je réaffirme mon souhait d'accueillir de nouveaux EPR à Tricastin, où tout un bassin d'emploi est prêt à se retrousser les manches pour participer à cette nouvelle aventure nucléaire. Nous en prenons conscience, les besoins en main-d'oeuvre qualifiée sont immenses

2022. S'agissant des ressources humaines, l'enjeu est considérable. Depuis 2020, 200 millions d'euros ont été consacrés à la formation dans cette filière. Dans notre région, nous anticipons aussi ces bouleversements. Un centre de formation aux métiers du nucléaire ouvrira ses portes en septembre 2023 à la Voulte-sur-Rhône, en Ardèche, en bordure de la Drôme. Je fais ici un clin d'oeil à mes collègues ardéchois, Mathieu Darnaud et Anne Ventalon. Ce centre devrait accueillir quatre-vingts élèves chaque année. Il leur permettra de se former aux différents métiers dont a besoin l'industrie nucléaire, comme la chaudronnerie, la soudure, l'usinage ou encore l'électricité. Un centre de formation d'autant plus nécessaire que ces métiers de techniciens et d'opérateurs ne sont pas suffisamment pourvus dans la filière, contrairement aux postes d'ingénieurs. Pour conclure mes chers collègues, en attendant de nous exprimer sur notre trajectoire énergétique, ce projet de loi sera essentiel pour accélérer, actualiser et dépoussiérer des procédures qui, pour certaines d'entre elles, datent de cinquante ans. Alors, mes chers collègues, votons ce projet de loi, rien que ce projet de loi, tout ce projet de loi

Le contexte, c'est celui de cinq années de désintérêt, de tergiversations au plus haut niveau de l'État, débouchant en février 2022 sur une décision de commande ferme de six EPR 2 et de mise à l'étude de huit unités supplémentaires, avec l'espoir d'une hypothétique mise en service, dans le meilleur des cas, en 2035, et sans avoir lancé de débat ou de consultation, un tant soit peu démocratiques, avec les premiers concernés : nos compatriotes. Pendant des années, nous avons sollicité, sans cesse, les gouvernements, les uns après les autres, afin d'engager ce débat avec les Français et, au Parlement, avec vous. Nous vous avons interpellée, madame la ministre, au sujet de la nécessité de prendre le temps d'avoir un débat approfondi sur le mix énergétique, qui doit évoluer au regard de l'indispensable sortie des énergies fossiles. Sans cesse, nous avons rappelé la situation alarmante d'EDF et attiré l'attention sur la crise de l'énergie que nous voyions se développer bien avant la crise géopolitique européenne actuelle.

Dans le cadre de quelle stratégie sommes-nous ? Avec quels moyens financiers ? Pour servir quels objectifs de souveraineté industrielle, dans l'intérêt premier des consommateurs aussi bien particuliers, professionnels qu'industriels ? Sur la base de quelles propositions françaises de réforme du marché européen ? Un marché qui a démontré son inadéquation avec les intérêts stratégiques des États membres et de l'Union européenne.

Sans débat de fond entre nous, portant sur ce que pourrait ou devrait être le mix énergétique, la majorité sénatoriale a élargi le périmètre du projet de loi initialement consacré à la simplification des procédures de délivrance des autorisations. Nous nous sommes opposés à ce changement de périmètre. Pourquoi ? Parce que ce débat ne peut pas être traité à la légère, au Parlement, au détour- et en quelques heures de discussion -d'un texte qui ne lui est pas entièrement consacré et qui n'a pas été préparé dans ce

et doivent pouvoir discuter des politiques énergétiques comme climatiques qui conditionneront la durabilité, si ce n'est la viabilité, du monde de demain. du trop peu de considération- c'est un euphémisme -accordée à la Convention citoyenne pour le climat, nous devons respecter les débats en cours,

Respecter la dimension consultative ou participative de notre démocratie ne nous permet pas d'anticiper le contenu de la future loi quinquennale, examinée par le Parlement en 2023. Le mix devra résulter d'un optimum combinant les différents modes de production disponibles, tout en tenant compte de leurs divers effets spécifiques. Nous n'écartons aucun moyen de production décarboné. Dans une perspective d'emplois et de souveraineté nationale, nous devrons nous donner l'objectif de disposer de filières industrielles implantées dans nos territoires. La formation et la reconnaissance des métiers devront être notre priorité ; cela pour chaque mode de production.

En considérant ces différents aspects, soyons réalistes et rationnels afin d'adopter une position politique éclairée, dont les effets seront majeurs à long terme. C'est la position de principe du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Quant au débat, l'ensemble de nos amendements tendant au rétablissement du périmètre initial ont été rejetés. Nous avons aussi voulu porter le débat sur des points de vigilance qui méritent l'attention. Il s'agit de ceux qui sont relatifs à la nécessaire prise en compte des aléas climatiques extrêmes- ressource en eau, trait de côte, inondations, etc. -, autant de sujets qui, avec d'autres, conditionneront la performance et la sécurité du parc de production nucléaire dans les décennies à venir.

des conséquences des procédures dérogatoires instaurées par ce texte, je soulignerai deux avancées issues de nos propositions. La première, c'est le renforcement du dialogue avec les exécutifs locaux en amont de la mise en oeuvre des procédures dérogatoires de mise en compatibilité des documents d'urbanisme.

permettra de gagner une année, deux au mieux, alors que le pays en a perdu cinq pour des installations industrielles dont la durée de vie pourrait être de soixante ans ou plus. En conséquence, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'abstiendra.

puisqu'il a toujours fallu intervenir pour faire émerger un semblant de concurrence. Et quelle concurrence ! Les fournisseurs alternatifs sont dopés aux aides d'État indirectes et propulsés par l'assèchement organisé de l'opérateur historique, EDF. Au sein du marché européen de l'électricité,

un fiasco pour les usagers, pour l'innovation, pour l'investissement et pour le développement des énergies décarbonées ! Cette situation, personne ne peut l'ignorer tant la crise l'a rendue visible les collectivités, les entreprises, les artisans, les commerçants, les particuliers, nul n'est épargné. Mais un choc n'est jamais une fatalité. Lorsque l'on prend la mesure de ce qui se produit

les sensibilités politiques sont loin d'être les mêmes, mais tous vous ont reproché la méthode avec laquelle vous avez abordé le sujet. Près de six mois avant la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie,

Madame la ministre, la filière nucléaire a souffert non pas des délais administratifs, mais des atermoiements des gouvernements successifs et de la volonté de mettre fin à cette filière. Quant à nous, communistes, nous soutenons le développement du nucléaire comme celui des énergies renouvelables, mais à deux conditions : démocratie et sécurité.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la situation du mix énergétique français est désormais

dans l'urgence, bien sûr ... Face aux multiples enjeux qui s'imposent à nous- la souveraineté énergétique, la baisse programmée de la consommation d'énergies fossiles, la nécessité de développer une énergie bas-carbone et, bien sûr, une plus grande efficacité énergétique -, le nucléaire doit être le fer de lance de la politique énergétique française pour les trente années à venir. Nous n'avons pas le choix qu'en construisant un mix énergétique alliant un nucléaire pilotable à des énergies renouvelables diversifiées et compétitives que nous pourrons envisager un avenir plus serein pour nos concitoyens, pour nos entreprises et pour notre planète.

Je ne m'attarderai pas trop longuement sur le joyeux désordre qui règne dans le calendrier parlementaire de la politique énergétique. Désormais, à chaque saison son projet de loi énergétique : l'automne nous a offert les énergies renouvelables ; l'hiver, le nucléaire ; le début de l'été nous verra examiner une loi de programmation aux contours complètement inconnus. Cette saisonnalité regrettable conduit notre politique énergétique à être au mieux illisible, au pire incohérente. Je ne reviendrai pas non plus dans le détail sur les actes manqués de ce texte, d'une technicité rare et au caractère politique limité, voire inexistant.

je ne m'arrêterai pas non plus longuement sur les questions soulevées quant à l'avenir de notre capacité de production électronucléaire. Selon RTE, notre mix énergétique devra être composé à 55 % d'électricité, contre 25 % actuellement.

inévitablement les réacteurs construits dans les années 1970 et 1980 fermeront. Mes chers collègues, vous l'avez compris, le compte n'y est pas. Nous devons donc être bien plus ambitieux afin de relever ce défi. Je souhaite néanmoins revenir sur le travail sénatorial de fond et de qualité mené à partir du projet de loi initial, travail qui a permis de consolider l'assise juridique du nucléaire existant, ainsi que le cadre des projets à venir. Je salue également l'excellent travail de nos rapporteurs,

Je souhaite relever quelques apports essentiels issus de leurs travaux, notamment la suppression par le Sénat de l'objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici à 2035.

disposition permettra de doter le nucléaire d'une vision stratégique plus claire et de long terme, et concourra à l'attractivité de la filière, qui est essentielle pour donner envie à nos jeunes de suivre les formations nécessaires à la relance du nucléaire. Autre point positif : la meilleure prise en compte de l'avis des collectivités territoriales dans la mise en compatibilité des documents d'urbanisme lorsqu'un projet de réacteur est à l'étude. Cette demande venait de nos territoires, c'est désormais chose faite et cela constitue un véritable pas en avant. Nous devons bâtir notre stratégie énergétique avec l'ensemble des acteurs concernés ; cela commence à l'échelon local. Enfin, la consolidation de la procédure de réexamen des réacteurs nucléaires au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement est inévitable, afin de garantir un bon

chers collègues, sous l'impulsion de nos rapporteurs, nous avons fait évoluer ce texte technique afin de faciliter concrètement la construction de futurs réacteurs. L'année 2023 doit être celle

des paroles aux actes, sans éluder, bien sûr, les questions essentielles d'approvisionnement en uranium, de gestion des déchets, de sûreté et de recherche et développement.

Mes chers collègues, si nous sommes actuellement confrontés à une crise économique importante et à une inflation galopante, c'est en grande partie parce qu'un certain nombre de responsables politiques ont torpillé le programme nucléaire français.

Acte est donné de cette demande. Pour l'examen de ce texte, nous pourrions prévoir une discussion générale de 45 minutes. Par ailleurs, le délai limite de dépôt des amendements de séance serait fixé au lundi 30 janvier à 12 heures. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle la désignation des dix-neuf membres de la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française, ainsi que des vingt et un membres de la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire en France. En application des articles 8 et 8 , alinéa 5, du règlement du Sénat, les listes de candidats remises par les groupes politiques ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle, en application de l'article 16 , alinéa 2, du règlement, la proposition de création d'une commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires. Je soumets cette proposition au Sénat. Il n'y a pas d'opposition ? ? ... Il en est ainsi décidé. Conformément à la décision de la conférence des présidents, la désignation des 37 membres de cette commission spéciale aura lieu en séance publique mercredi 1 février.

17, 4 et 5, ainsi que l'amendement portant article additionnel après l'article 4, soient examinés en priorité avant l'article 3 que les articles 9 à 11, ainsi que les amendements portant articles additionnels s'y rapportant, soient examinés avant l'article 8 ; enfin, que l'article 18 soit examiné avant l'article 12.

l'accueil du monde entier, autour des valeurs de l'olympisme : l'excellence, l'amitié, le respect ; des performances qui ont inspiré les générations futures et les ont poussées à aller, à leur tour, plus vite, plus haut, plus fort ; des infrastructures durablement améliorées et une première reconnaissance du sport féminin voilà ce que les Jeux de 1924 avaient légué à la France. C'était il y a presque cent ans. Chacun le sait, en réinventant les Jeux de l'ère moderne, Pierre de Coubertin portait le rêve d'un événement capable d'une influence positive sur le cours du monde ; ces compétitions ont su s'affirmer au fil du temps comme d'exceptionnels moments de rapprochement entre les peuples. Les Jeux ont été à l'origine d'exploits sportifs fascinants, d'émotions collectives à nulle autre pareille. Pour les pays hôtes, organiser et réussir les Jeux est donc un honneur conquis de haute lutte, une formidable opportunité, mais aussi, chacun le mesure, un immense défi. Aujourd'hui, la France retrouve les jeux Olympiques pour la première fois depuis un siècle et accueille les jeux Paralympiques pour la première fois de son histoire. C'est à Lausanne, il y a cinq ans, sous l'égide du Président de la République, que le rêve olympique et paralympique français est devenu vraisemblable ; c'est à Lima qu'il a pris réalité. La délégation française a forgé alors cet « esprit de Lima », un esprit d'unité qui a permis de poser les fondations des Jeux de Paris 2024 ; un esprit que nous ferons vivre.

de la Première ministre. Avec beaucoup de gratitude, je tiens à remercier ceux qui ont été les pionniers de cette conquête olympique collective. Je me tourne notamment vers vous, cher Patrick Kanner, je salue également les sénateurs qui contribuent à cette aventure collective et ceux qui, plus largement, portent, parfois depuis longtemps, la volonté de voir le sport mieux installé au coeur de notre société. À ce titre, je tiens tout particulièrement à remercier la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, ainsi que son président, Laurent Lafon, pour sa vision et pour nos échanges, aussi exigeants que constructifs.

S'y ajoute l'ensemble des ministères concernés, tous mobilisés et coordonnés par la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques, dirigée par le préfet Michel Cadot.

publiques et privées. J'ai l'habitude de dire que réussir les Jeux, c'est réunir un quatuor d'exigences : l'organisation la plus irréprochable possible ; des athlètes au meilleur de leur performance

qui hantent encore certaines rues d'Athènes et de Rio. L'exemplarité écologique : elle s'exprimera notamment au travers d'une division par deux des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux éditions précédentes. La maîtrise des budgets : en dépit du contexte d'inflation que chacun connaît,

qu'il nous reste à adopter afin d'aller au bout de nos engagements et de nos besoins opérationnels pour la livraison et le bon déroulement des Jeux. C'est tout l'objet du projet de loi que j'ai aujourd'hui l'honneur de défendre devant vous. Permettez-moi d'en exposer les principaux objectifs. Il s'agit, d'abord, de soigner et de porter secours. Il nous revient de créer, le temps des Jeux, un centre de santé au sein du village olympique et paralympique pour les athlètes et les personnes accréditées. Ce centre sera géré, dans un cadre simplifié, par

cette polyclinique. Nous comptons aussi étendre la liste des organismes habilités à former aux premiers secours, au-delà des associations agréées de sécurité civile. deuxième objectif de ce texte -promouvoir un sport sans dopage. Par ce texte, nous entendons maintenir la France à l'avant-garde de la lutte contre le dopage, où, en leur temps, mes prédécesseurs Marie-Georges Buffet, Jean-François Lamour et Valérie Fourneyron ont su la placer. Il nous faut rester à ce niveau d'excellence et continuer de répondre à nos obligations internationales en la matière, édictées par l'Agence mondiale antidopage et découlant de la convention de l'Unesco, ratifiée par le Parlement.

ouvrir la possibilité de réaliser des analyses génétiques, comme cela a été fait à Pékin et à Tokyo, afin de déceler les fraudes qui ne peuvent l'être d'aucune autre façon et, ainsi, éviter qu'une faille, un point de fuite, dans notre édifice ne vienne en ruiner la crédibilité tout entière.

pour des situations et des finalités limitativement énumérées ; mise en oeuvre au moyen d'échantillons anonymisés et promptement détruits, ne permettant ni identification, ni sélection, ni profilage des sportifs concernés. Nous avons ainsi veillé à concilier au mieux les impératifs de l'éthique et de l'intégrité sportives, dans le respect de nos obligations internationales.

des enceintes sportives, avec quatre cérémonies d'ouverture et de clôture, le relais de la flamme, mais également la préservation de l'ordre public et la prévention de la délinquance aux abords de tous nos sites, la cybersécurité, ou encore la gestion efficace des flux de personnes, depuis l'arrivée sur le territoire national jusqu'à nos métros, nos bus et nos RER. de ce projet de loi, nous entendons donc nous doter de moyens renforcés pour détecter plus rapidement et plus facilement, par la vidéoprotection, les risques graves- mouvements de foule, colis suspects, goulets d'étranglement dans les transports ... -, mais aussi améliorer et fluidifier le contrôle à l'entrée des sites de compétition et de célébration. Il importe de mieux coordonner les équipes mobilisées pour la sécurité dans les transports et d'assurer une unité de commandement des forces de sécurité pendant la période des Jeux. Là aussi, nous avons entendu les questions posées sur la nature de certains dispositifs, comme le traitement par algorithme des images de vidéoprotection, qui continue de susciter des interrogations sur certaines travées de cet hémicycle. nous souhaitons souligner que les très nombreuses garanties mises en place dans le cadre de cette expérimentation nous aideront à être au rendez-vous de la sécurité des Jeux tout en préservant les droits et les libertés de nos concitoyens, en parfaite conformité avec le droit européen de la protection des données.

Je salue, à cet égard, le travail réalisé par les deux commissions du Sénat qui ont analysé ces incidents, puis recommandé un ensemble d'améliorations dont nous avons tenu compte dans ce projet Ainsi, nous souhaitons renforcer les sanctions individuelles prononcées par le juge judiciaire en cas d'entrée par force ou par fraude dans les enceintes, ou d'intrusion sans motif légitime sur l'aire de compétition. De même, il vous est proposé de rendre systématiques les interdictions judiciaires de stade pour les infractions pénales les plus graves, par exemple l'introduction d'objets susceptibles de constituer une arme, les jets de projectiles, la provocation à la haine ou à la violence, ou encore l'incitation à la discrimination.

de moins de 250 taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) à plus de 1 000. Pour cela, nous souhaitons permettre à titre expérimental au préfet de police de délivrer de nouvelles licences de taxi PMR dans des conditions simplifiées. cinquième objectif est de favoriser le potentiel économique dans les territoires. À ce titre, ce projet de loi doit d'abord nous permettre de respecter les engagements du contrat de ville hôte en matière publicitaire vis-à-vis des partenaires des Jeux, lors du relais de la flamme et du compte à rebours, tout en les conciliant avec l'exigence de protection de l'environnement. L'activité commerçante doit aussi être en mesure de répondre à l'afflux de touristes, de spectateurs et de travailleurs. À cette fin, il vous est proposé de permettre aux préfets

à l'avenir de la Solideo, appelée à se rapprocher de Grand Paris Aménagement. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, l'essentiel des dispositions que nous vous soumettons. Nous avons veillé à définir, de manière claire et transparente, celles qui sont limitées

pour la qualité de leurs analyses, de nos échanges et de leurs propositions sur ce texte. Je veux aussi saluer les apports des travaux en commission : j'ai en particulier à l'esprit l'amélioration du cadre envisagé pour les analyses génétiques antidopage, le déploiement d'une billetterie nominative, dématérialisée et infalsifiable pour certaines compétitions sportives, ou encore l'ajustement le plus proportionné possible à la gravité des faits des mesures de lutte contre les violences dans les stades. Tout au long de nos débats, je serai à votre écoute, avec la volonté d'améliorer ce projet de loi

C'est donc dans la fidélité à cet esprit d'innovation que les Jeux de Paris 2024 vont dessiner une nouvelle référence olympique. Ils offriront une occasion unique de faire de faire rayonner la France, une France ouverte sur le monde, audacieuse et responsable, assumant ses idéaux universels et son amour pour le sport. La parole

Les Olympiades sont plus qu'un simple rendez-vous sportif : il s'agit d'un moment de cohésion nationale et de fraternité humaine. C'est également une vitrine pour le pays hôte : la France exposera aux yeux du monde le savoir-faire français et une certaine façon de célébrer l'esprit olympique, par le mérite, la maîtrise de soi, le dépassement. Ce sera surtout un événement d'une ampleur exceptionnelle. D'un point de vue sportif, d'abord : 10 500 athlètes de 32 disciplines différentes se mesureront lors de 549 épreuves. En matière d'organisation, ensuite : les compétitions se dérouleront dans 37 sites olympiques, jusqu'en Polynésie pour le surf, et mobiliseront 63 collectivités hôtes et plus de 40 000 bénévoles. Enfin, d'un point de vue événementiel, cette fête réunira 13,5 millions de spectateurs, 20 000 journalistes accrédités et quatre milliards de téléspectateurs dans le monde entier. Fait inédit, la cérémonie d'ouverture prendra place le long de la Seine, sur six kilomètres, du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna, où se dérouleront les spectacles et les cérémonies protocolaires. Ce sera la première fois qu'un tel événement se tient en dehors d'un stade fermé. Cette innovation, qui devrait réunir 600 000 spectateurs, représente aussi un défi en termes de sécurité. Cette grande fête populaire et sportive focalisera l'attention du monde entier ; elle impose une organisation exemplaire. Livrer les Livrer les équipements dans les temps, faire monter en puissance les capacités de transport, coordonner les différents acteurs et prévoir une organisation de la sécurité à la hauteur de l'événement constituent autant de défis qui devront être relevés d'ici à juillet 2024

Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport rendu il y a quelques jours, « la phase de planification stratégique des Jeux de Paris 2024 s'est globalement bien déroulée ». Il convient, désormais, de passer à la phase de déclinaison opérationnelle. Tel est l'objet de ce nouveau projet de loi soumis à notre examen.

Si toutes ces dispositions, souvent techniques, sont nécessaires à la réussite des jeux Olympiques, deux dispositifs nouveaux soulèvent cependant l'épineuse question du juste équilibre entre la recherche d'efficacité et la garantie des droits et libertés individuelles, que ce soit en matière de lutte contre le dopage ou de sécurisation des jeux. La France s'est engagée avec force, depuis les années 1990, dans la lutte contre le dopage, essentielle pour assurer l'équité entre les sportifs et garantir leur santé. Afin d'obtenir l'organisation des Jeux de 2024, la France a promis de compléter son arsenal de mesures antidopage par l'introduction des tests génétiques, conformément aux engagements internationaux qu'elle Paradoxalement, alors que l'introduction du recours aux tests génétiques assure la mise en conformité du droit français avec le code mondial antidopage, l'article 4 du projet de loi, dans sa version initiale, ne devait s'appliquer que jusqu'au 31 décembre 2024. comment accepter que les sportifs français ne puissent pas être soumis aux tests génétiques en France alors qu'ils y sont soumis partout ailleurs ? En effet, ces tests sont aujourd'hui les seuls à permettre de confirmer la manipulation d'échantillons, d'écarter une suspicion de transfusion de sang homologue, de vérifier l'inexistence d'une mutation génétique rare conduisant à un taux d'érythropoïétine (EPO) supérieur à la moyenne, ou de détecter les manipulations génétiques qui permettent d'augmenter la performance. C'est pourquoi la commission des lois a adopté un amendement tendant à réécrire l'article 4 de manière à inscrire dans le code du sport la possibilité de recourir aux tests génétiques pour les deux premières finalités

posait des difficultés techniques et n'assortissait pas l'ensemble des tests des mêmes garanties. C'est pourquoi je vous proposerai de pérenniser l'ensemble de ces tests tout en renforçant les garanties afférentes.

Surtout, l'ampleur des jeux Olympiques et Paralympiques impose de se doter d'une organisation irréprochable en matière de sécurité, d'autant que la menace terroriste est toujours élevée en France. À cela s'ajoutent deux risques majeurs : le risque cyber et le risque sanitaire. Par ailleurs, la sécurisation de la cérémonie d'ouverture en plein air complexifie la tâche. Les premières estimations indiquent que les Jeux nécessitent la mobilisation de moyens quotidiens humains et matériels substantiels 22 000 et 33 000 agents de sécurité privés, dont le recrutement pose d'ailleurs quelques difficultés, et 45 000 agents publics- forces de sécurité intérieure et armée. L'acceptabilité des Jeux implique en outre qu'un équilibre soit trouvé entre les missions de sécurité liées aux Jeux et la permanence des autres mesures sur le reste du territoire. L'utilisation des images prises par les caméras de vidéoprotection ou les drones doit être renforcée pour aider les forces de l'ordre à sécuriser les espaces publics ; trois articles y concourent.

L'expérimentation de l'utilisation de la vidéoprotection « intelligente » ou « augmentée », inscrite à l'article 7, est une innovation majeure, mais elle soulève de nombreuses interrogations en matière de libertés publiques, qu'il convient de mettre en balance avec les avancées opérationnelles permises par un tel dispositif, notamment pour les Jeux. Le traitement par des algorithmes des images captées permettra de détecter et de signaler des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes. Il constituera un outil d'aide à la décision pour les forces de sécurité, qui pourront ainsi se concentrer sur l'action.

Réécrit après les avis du Conseil d'État et de la Cnil, l'article 7 instaure de nombreuses garanties à chaque étape de la mise en oeuvre de ce dispositif. La commission des lois du Sénat a considéré que ces garanties assuraient un équilibre satisfaisant entre la protection des droits et libertés et la plus grande opérationnalité en matière de sécurité. Elle a d'ailleurs souhaité sécuriser cette procédure en renforçant le contrôle assuré par la Cnil, tant dans la mise en oeuvre du traitement que dans le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Enfin, le criblage des fan zones et de tous les participants, ainsi que l'autorisation du recours aux scanners corporels à ondes millimétriques pour les gestionnaires d'enceintes sportives qui le souhaitent, assureront eux aussi une meilleure sécurisation des grands événements accueillis par la France.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales s'est vu déléguer l'examen des dispositions du présent texte qui concernent la santé et le travail. L'article 1 prévoit la création de la polyclinique olympique et paralympique, sous la forme d'un centre de santé au statut aménagé. La structure, qui sera gérée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, vise à mettre à la disposition des seuls athlètes et personnes accréditées une offre de soins de premier recours. Outre un encadrement composé de salariés de l'AP-HP, le fonctionnement du centre reposera sur des praticiens volontaires olympiques et paralympiques. Au pic d'activité, ceux-ci devraient être au nombre de 193, dont 36 médecins, 28 masseurs-kinésithérapeutes et 14 infirmiers. Trois principales dérogations ont été identifiées comme nécessaires au fonctionnement de ce centre de santé, afin de clarifier le public spécifique restreint auquel la polyclinique s'adresse et de prévoir la gratuité des prestations réalisées ainsi que la présence d'une pharmacie hospitalière. Le même article 1 simplifie également différentes procédures relatives au projet de santé, ou encore à l'installation d'équipements d'imagerie. La commission des affaires sociales a soutenu le dispositif proposé et a veillé à préciser le statut dérogatoire de la polyclinique. L'article 2 complète l'article 1 quant à l'organisation d'une offre de soins spécifique aux Jeux, en autorisant l'exercice de leur profession à trois grandes catégories de professionnels de santé qui seraient mobilisés pour l'événement, mais ne justifieraient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France.

Enfin, l'article 2 autorise l'exercice de leur profession aux professionnels de santé étrangers qui pourraient participer à l'activité de la polyclinique en tant que volontaires, selon une procédure qui reste toutefois à établir avec le Conseil La commission des affaires sociales a approuvé ces dispositions. Elle a également approuvé la création, à l'article 17, d'une dérogation au repos dominical pour les commerces de détail situés dans les communes où auront lieu les compétitions, ainsi que dans les communes limitrophes et à proximité. Les très nombreux visiteurs attendus pendant les Jeux doivent être accueillis dans les meilleures conditions, d'autant que les besoins du public seront source de développement économique. Cette dérogation est assortie de garanties pour les salariés : parmi eux, seuls les volontaires travailleront le dimanche ; ils bénéficieront d'une rémunération doublée et de repos compensateurs. Elle s'ajoutera aux dérogations déjà existantes, comme les dimanches du maire ou les ouvertures en zone touristique, afin de s'adapter aux besoins exceptionnels liés aux jeux Olympiques et Paralympiques. Compte tenu des nombreuses demandes de dérogations attendues, des besoins du public déjà prévisibles et du caractère bien circonscrit de la mesure, notre commission a simplifié la procédure d'autorisation préfectorale, afin que le préfet puisse d'emblée autoriser un ou plusieurs établissements à déroger au repos dominical, au lieu de procéder par autorisation individuelle, puis par arrêté d'extension. un mot de l'article 4, dont la commission des affaires sociales s'est saisie pour avis. Cet article complète l'arsenal de la lutte antidopage en autorisant l'examen des caractéristiques génétiques de rechercher quatre méthodes possibles d'amélioration des performances. Il prévoit également l'orientation du sportif vers une consultation adaptée lorsqu'un tel examen entraîne la découverte incidente d'une caractéristique responsable d'une possible affection.

comme cela a été rappelé, ce projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 constitue probablement la dernière occasion d'adapter notre droit de manière à assurer la bonne tenue de cet événement. Il constitue également une première opportunité de tirer les conséquences des événements survenus au Stade de France le 28 mai 2022, qui ont vu de très nombreux délinquants forcer l'entrée du stade et plusieurs milliers de fraudeurs tenter de s'introduire avec des billets falsifiés.

au moment où plusieurs centaines de milliers de spectateurs s'apprêtent à nous rendre visite, en 2023 et en 2024, pour assister à la Coupe du monde La commission de la culture, qui s'est vue déléguer au fond l'examen des articles 12, 13 et 14, a souhaité tirer toutes les conséquences de ces événements en modifiant le texte selon deux axes.

qui tentent de s'introduire dans les enceintes sportives ou sur les aires de compétition. Notre commission a créé à cette fin une nouvelle amende délictuelle, de manière à renforcer l'effet dissuasif de ces dispositions tout en respectant le principe de proportionnalité des peines. Notre commission a émis un avis défavorable sur plusieurs amendements visant à réduire les peines encourues par les délinquants qui cherchent à entrer de force dans les stades, à ne pas condamner les activistes qui interrompent les retransmissions sportives pour imposer leur message politique, ou encore à rendre inopérant le dispositif des interdictions de stade. de stade. Je constate que la volonté de lutter contre les violences de toute nature qui prolifèrent dans nos stades ne fait pas consensus. Je le regrette d'autant plus que nous avons observé, ces derniers mois, une augmentation des violences dans le sport au sens large ; il ne me semble pas envisageable de baisser la garde à quelques mois du début des jeux Olympiques et Paralympiques. Je veux enfin rappeler la nécessité, pour chacun d'entre nous, de concourir le mieux possible au succès de ces jeux Olympiques et Paralympiques. Pour le Parlement, cela signifie au moins deux choses.

En second lieu, il nous revient de veiller aux équilibres budgétaires de cet événement. Tel est le sens de notre amendement visant à faire remettre au Parlement un rapport d'étape dressant un bilan des Jeux avant le 1 octobre 2025. Nos échanges avec la Cour ont permis d'établir le caractère indispensable de ce rendez-vous qui, bien entendu, n'obérera en rien les travaux que celle-ci mènera d'ici à 2026 pour réaliser un bilan financier définitif de cet événement. Il me paraît toutefois essentiel que les Français sachent que leurs élus veillent au respect du budget des Jeux, compte tenu de la garantie financière apportée par l'État. Je terminerai en remerciant Mme la rapporteure Agnès Canayer,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la Charte olympique, « le but de l'Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine Dans notre monde globalisé, le sport a ce pouvoir unique de rassembler les peuples. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste ne peut que souscrire à l'esprit des jeux Olympiques. Mes chers collègues, mon groupe émettra des critiques, mais en aucun cas nous ne dévaluerons l'importance du sport, qui est l'un des quelques domaines universels de l'activité humaine. Des règles, Des règles, mais également des valeurs, universelles l'encadrent- celles du fair-play, du respect et de l'amitié -, qui sont reconnues dans le monde entier. Notre groupe reconnaît et soutient le pouvoir rassembleur, le pouvoir d'intégration du sport. nous ne pouvons que regretter et dénoncer un texte hautement sécuritaire qui porte mal son nom, puisqu'il nous parle, hélas ! moins de sport que de sécurité. Le groupe CRCE considère que la devise olympique « Plus vite, plus haut, plus fort » est ici détournée pour un « plus vite, plus haut, plus fort » de sécurité et d'atteinte au droit à la vie privée, protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de cette même déclaration. Ce projet de loi- j'ai déjà eu l'occasion de le dire -est un cheval de Troie, tant les dispositions attentatoires aux libertés et aux droits fondamentaux qu'il comporte seront susceptibles d'être pérennisées- c'est déjà le cas pour onze d'entre elles. elles. Nous dénonçons un projet de loi porteur de graves atteintes à des libertés constitutionnellement garanties. Dans ces conditions, mon groupe se doit de tirer la sonnette d'alarme. Nous ne laisserons pas passer de telles atteintes, qui gâcheraient la fête.

À titre d'exemple, la Seine-Saint-Denis accueillera le village olympique en 2024. En tant que sénatrice de ce département, je suis inquiète. Le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des champions, en mai 2022, a mis en lumière les carences de la France pour assurer la sécurité d'un événement sportif majeur. Pourtant, face face à cet enjeu dont vous reconnaissez l'importance, vous nous proposez de recourir à des entreprises privées. Nous dénonçons cette réponse, qui n'est pas à la hauteur de l'ambition nécessaire. Oui, mes chers collègues, le recours aux 22 000 à 33 000 agents de sécurité privée demandés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques pour encadrer les Jeux confirme la tendance à l'intégration de la sécurité privée en tant que force de police institutionnalisée et bras armé de l'État.

de la sécurité privée dissimule également la marchandisation de la sécurité publique et la délégation de missions de service public à des entreprises qui ont pour unique finalité la recherche de la rente, une finalité bien éloignée des fonctions régaliennes de l'État.

Lopmi. Nous regrettons que la gestion sécuritaire des Jeux se traduise également par les opérations antidélinquance menées depuis novembre 2022 et qui continueront jusqu'aux Jeux. Aujourd'hui, deux opérations antidélinquance d'envergure sont menées chaque jour à Paris et en Seine-Saint-Denis, auxquelles s'ajoutent deux opérations dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, sans compter les initiatives de moindre ampleur pluriquotidiennes. Entre le 7 et le 27 novembre, 235 de ces opérations ont été conduites, pour une cinquantaine de gardes à vue.

». Mon groupe s'oppose tout aussi fermement à la légalisation de la vidéosurveillance algorithmique portée par ce projet de loi. La détection par logiciel d'événements et de comportements dits « suspects » portera, une nouvelle fois, une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et à la liberté d'aller et venir des participants. Cette légalisation sera l'occasion, pour les entreprises françaises, de montrer leur savoir-faire en matière de répression et, pour le Gouvernement, de déployer une technologie encore illégale, mais dont l'offre commerciale est pourtant

de ce texte, tout aussi important. Alors que l'Assemblée nationale s'apprête à entamer l'examen de la réforme des retraites, le présent projet de loi prévoit un recul scandaleux de la limite d'âge des fonctionnaires occupant des emplois participant directement à l'organisation des Jeux, « au nom au nom de l'intérêt du service », et ce jusqu'au 31 décembre 2024. Dans la même veine, l'ouverture le dimanche des commerces de vente dans les communes des sites de compétition et à proximité remet en cause le principe du repos dominical et porte atteinte au droit fondamental à la vie privée et familiale.

Le texte autorise donc, pour le temps des Jeux, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par ses empreintes génétiques afin d'améliorer les contrôles antidopage. Si cette transposition d'une norme internationale encadrant le contrôle antidopage est nécessaire au déroulement des Jeux, mais aussi de la Coupe du monde de rugby, la Cnil et la Ligue des droits de l'homme dénoncent en des tests particulièrement intrusifs, qui dérogent de façon importante aux principes encadrant actuellement les analyses génétiques dans le code civil paradoxalement temporaire de cette mesure qui sera appelée à se pérenniser, et ce alors même qu'elle déroge de manière disproportionnée à des dispositions du code civil. Enfin, que la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques pouvait représenter une formidable opportunité de modernisation et d'amélioration de la qualité du service du réseau francilien, se pose aujourd'hui la question de la capacité d'Île-de-France Mobilités à répondre au défi de la saturation. Alors que de nouvelles lignes de métro auraient dû être prêtes pour relier les différents sites olympiques et permettre le transport de 10 millions de personnes, seul le prolongement de la ligne 14 sera livré à temps. Les promesses de réponse aux besoins de mobilité générés par les Jeux au moyen de solutions décarbonées peineront à être tenues, et ce n'est pas la privatisation voulue par certains qui améliorerait la situation

et le droit au respect de la vie privée des usagers. En conclusion, mon groupe considère que ce projet de loi libéral et sécuritaire ne respecte pas le juste équilibre entre sécurité et protection des libertés et droits fondamentaux.

Nos collègues communistes souhaitent que l'examen de ce texte s'achève avant même d'avoir réellement débuté, jugeant qu'un certain nombre de ses dispositions sont attentatoires aux libertés publiques. Telle n'est pas la position d'abord, la tenue des jeux Olympiques est imminente ; des délais supplémentaires ne feraient que compliquer, voire rendre impossible, la tâche des organisateurs, qui attendent avec impatience le vote de ce texte final, complétant celui de 2018. Ensuite, nous devons tirer les conséquences des événements survenus au Stade de France le 28 mai

travail des rapporteurs, ne sont pas contraires à la Constitution. Nous estimons que la conciliation entre les exigences de protection des personnes durant les événements sportifs et de protection des libertés publiques, qui sont chères à notre assemblée La protection des données est suffisante et les différents dispositifs de sécurité instaurés sont encadrés dans leur champ comme dans leurs usages.

collègues, nous aurions vraiment aimé légiférer sur le sport- c'est suffisamment rare ! Nous aurions aimé légiférer pour que les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 se déroulent dans les meilleures conditions et qu'ils laissent un héritage à la hauteur des ambitions environnementales fixées à l'origine. Nous aurions adoré adoré jouer notre rôle de législateur pour vous accompagner, madame la ministre, dans l'organisation d'un événement auquel nous sommes attachés et dont nous partageons les valeurs, celles de l'olympisme. Nous aurions aussi aimé débattre sérieusement des conséquences de cet événement sur notre tissu de festivals et d'événements culturels. Nous aurions pu rassurer les milliers de professionnels qui voient leur saison de festivals menacée par des annonces verticales et autoritaires prises sans concertation. De tout cela, il n'y a rien, ou très peu, dans ce projet de loi. En revanche, au coeur de ce texte se sont glissées des innovations législatives hasardeuses qui n'ont rien à y faire. Par une manoeuvre d'opportunisme législatif, ce projet de loi s'est éloigné de son ambition initiale pour faire des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 2024 un laboratoire d'expériences sécuritaires. Le public, national ou international, devient, grâce à ce texte, le cobaye d'une fuite en avant expérimentale dans la technologie de surveillance. Comment en sommes-nous arrivés là ? Par quel cheminement politique est-on parvenu à la conclusion que l'événement sportif mondial le plus fédérateur ne pourrait être organisé sans le déploiement de technologies d'intelligence artificielle et d'algorithmes de surveillance ? il y a bien eu un rapport sénatorial sur ces technologies, mais des rapports du Sénat, on en connaît des dizaines qui n'ont pas eu pour destin d'être transformés en loi d'exception ou d'urgence. Non, il y a eu un événement déclencheur, un événement traumatisant il faut au moins cela pour aboutir à la réussite d'un bon cavalier législatif. Cet événement, on le connaît ; le monde entier le connaît, puisqu'il s'est déroulé en mondovision devant des centaines de millions de téléspectateurs, le 28 mai 2022, le soir de la finale de la Ligue des champions. La capacité de la France à organiser un grand événement sportif international a été, ce soir-là, sérieusement mise en doute. Les mensonges, manquements et approximations du ministre de l'intérieur comme du préfet de police ont été mis au jour, notamment par notre Haute Assemblée, lors de

effet, l'intelligence artificielle aurait-elle permis d'éviter la défaillance dans l'orientation des supporters anglais ? L'intelligence artificielle aurait-elle déconseillé l'usage immodéré des gaz lacrymogènes sur des supporters pacifiques ? L'intelligence artificielle aurait-elle tiré, en amont, les conclusions d'une grève touchant l'une des deux lignes de RER qui menaient au Stade de France ? En d'autres termes, l'intelligence artificielle aurait-elle fait mieux que les intelligences combinées du ministre Darmanin et du préfet Lallement ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, je ne le pense pas.

plus que prudente sur ces technologies, en indiquant qu'elles sont susceptibles d'affecter les garanties fondamentales apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et qu'il serait donc nécessaire de changer la loi changer la loi, et non expérimenter une nouvelle technologie au mépris de nos libertés publiques. Non, nos libertés publiques ne peuvent être sujettes à une approche expérimentale ! Non, nos libertés publiques n'ont pas à être le terrain de jeu des start-ups de la sécurité Non, nos libertés publiques comme nos données ne doivent pas être marchandées à la légère avec des apprentis sorciers sécuritaires ! Oui, nous avons besoin d'un débat approfondi et éclairé sur ce changement radical dans notre approche de l'espace public. Il a d'ailleurs lieu au niveau européen, mais n'a toujours pas abouti. Le fait même d'expérimenter cette technologie est une menace pour nos libertés publiques, pour notre organisation sociale et pour nos débats démocratiques. Certes, la promesse de cette technologie est simple : elle faciliterait la détection de situations permettant de présumer la commission d'infractions ou encore la survenue d'événements suspects ou potentiellement dangereux. Pour cela, elle traite en temps réel des milliers d'images de vidéosurveillance. Par « traiter », il faut comprendre qu'elle les confronte avec un certain nombre de critères préétablis. Afin que ce traitement soit pertinent, l'algorithme a besoin d'apprendre.

Paralympiques, offrent à ces sociétés : les Jeux deviennent l'occasion rêvée de nourrir la bête. L'enjeu réel est là. Il n'est pas dans l'assistance supposée de ces outils au moment de l'événement, madame la ministre ; il est dans l'incroyable masse de données que les start-ups qui auront décroché le marché pourront collecter lors de l'événement. Ne vous faites pas d'illusion sur les garde-fous qui ont été introduits dans cette loi. L'ensemble des données sont utiles à l'algorithme : croire qu'il sera possible d'effacer les données non pertinentes n'a pas de sens quand on parle d'« apprentissage machine ». Les moments durant lesquels il ne se passe rien sont tout aussi utiles que ceux où se déroulent les événements problématiques, ne serait-ce que pour apprendre à la machine à les distinguer. Vous n'y connaissez rien du tout ! L'expérimentation qui est proposée n'offre donc aucune garantie sur les droits et libertés des personnes pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que ces algorithmes ne sont ni contrôlables ni transparents. Aussi, nous aurons beau demander dans ce texte que le traitement des données soit « loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l'occurrence de biais et nous n'en aurons aucune garantie. Tel est le coeur du problème lorsqu'on légifère sur des algorithmes fermés et opaques. Le ministre de l'intérieur s'est montré très respectueux du cadre législatif, puisqu'il s'est engagé à ne pas utiliser de technologies qui n'auraient pas été légalisées au préalable.

Oui, le ministre de l'intérieur, celui-là même qui nous demande aujourd'hui de déployer ces technologies dans un cadre de confiance, s'est montré incapable de faire respecter la loi qui les encadre déjà très strictement ! Tout en ayant visiblement connaissance d'usages illégaux de technologies de surveillance, n'agit pas pour faire respecter nos libertés ! Quelles garanties avons-nous que toutes les données collectées lors des Jeux ne serviront pas à nourrir des algorithmes de surveillance, vendus par les sociétés qui les exploiteront pendant les Jeux à des régimes moins précautionneux en matière de libertés publiques ? Acceptez-vous, chers collègues, que la grande fête des jeux Olympiques serve à nourrir les équipements de répression des mouvements de révolte contre les tyrannies à l'autre bout du monde ? Mes chers collègues, comme vous, je suis attaché au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Comme vous, je souhaite que la centaine de milliers de spectateurs attendus passe un moment extraordinaire à vibrer à l'unisson des valeurs de l'olympisme. Mais nous devons nous garder de tout opportunisme sécuritaire. Les jeux Olympiques ne doivent pas nous laisser en héritage une société de la surveillance globale. C'est pourquoi je vous propose de rejeter ce texte, afin que la ministre des sports puisse en expurger les dispositions qui n'ont rien à voir avec l'événement et que nous puissions revenir rapidement à une réelle discussion sur les enjeux réels de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La parole

sont à mon sens tout à fait contestables et je m'efforcerai de le démontrer, point par point. Premièrement, vous contestez l'expérimentation portant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. vous, la création d'un cadre juridique nouveau autorisant l'usage de l'intelligence artificielle pour le traitement d'images de vidéosurveillance traduirait une volonté indéniable du Gouvernement de pérenniser ces expérimentations, au motif que cela cela s'appliquerait au-delà des seuls sites olympiques et pour une durée dépassant largement celle des Jeux. Permettez-moi de rappeler que le dispositif envisagé, qui s'inspire de celui qui est prévu dans la proposition de règlement européen sur les systèmes d'intelligence artificielle en cours d'élaboration, est assorti de nombreuses garanties. S'agissant de la temporalité, la proposition du Gouvernement d'expérimenter le dispositif jusqu'au 30 juin 2025 ne cache aucune volonté de pérennisation. D'abord, les traitements en question n'utiliseront aucun système d'identification biométrique ; ils ne traiteront aucune donnée biométrique et ne mettront en oeuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ensuite, la Cnil devra être régulièrement informée des conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation, qui fera l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme, fixé au 30 juin 2025. Par conséquent, si la durée de l'expérimentation excède la date de la fin des Jeux, à savoir le 8 septembre 2024, rien ne permet d'affirmer à ce jour que les dispositifs seront reconduits et encore moins sous quelles modalités. S'agissant des lieux concernés par l'expérimentation, il semble justifié de ne pas limiter le périmètre aux sites olympiques : au vu de l'ampleur de l'événement et du nombre de visiteurs, sécuriser les Jeux n'a rien d'évident. Le dispositif concernerait les abords immédiats, ce qui inclut notamment le périmètre des sites d'interconnexion où les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP affectés au centre de la préfecture de police de Paris pourraient intervenir ponctuellement. Le Conseil d'État l'a souligné : l'expérimentation est destinée à rendre plus plus efficace le maintien de l'ordre pour un événement d'une telle ampleur et elle sera bel et bien limitée dans le temps et dans l'espace. C'est inexact ! Deuxièmement, vous évoquez un renforcement injustifié des interdictions de stade et des sanctions en cas de pénétration dans une enceinte sportive, disposition qui viserait tout particulièrement les militants écologistes. Cher Thomas Dossus, rassurez-vous : aucune mesure contenue dans ce projet de loi ne vise les militants écologistes ! Vous n'êtes pas sans savoir que, le 28 mai 2022, date de la finale des incidents se sont produits au Stade de France, notamment parce que des personnes ont pénétré ou ont tenté de pénétrer dans le stade par force ou par fraude. L'article 12 de ce texte, créant les deux nouveaux délits, vise précisément à sanctionner ces personnes qui s'introduisent dans une enceinte sportive sans détenir de billet

Une telle situation juridique ne peut subsister et nous devons renforcer la dissuasion afin d'éviter ce type d'incident nuisible au public, aux athlètes et à la France en tant que pays organisateur. Enfin, pour ce qui est de la pénétration ou du maintien sans motif légitime d'une personne dans l'aire de compétition d'une enceinte sportive, je rappelle que le but recherché est de sanctionner les personnes qui troublent la tranquillité de la manifestation sportive, par une amende de 7 500 euros, lorsque l'acte est commis en réunion ou en récidive. En dehors de ces deux cas, la sanction sera celle d'une contravention de cinquième classe, à savoir une amende maximale de 1 500 euros. Actuellement, l'entrée sur l'aire de jeu d'un stade ne peut être incriminée que dans deux situations : lorsqu'elle trouble le déroulement de la compétition ou lorsqu'elle porte atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Encore une fois, il s'agit de prévenir, autant autant que faire se peut, des incidents de ce genre, qui troubleraient la fête, le bien-être des sportifs et la tranquillité du public, sans occulter le principe de proportionnalité des peines. Troisièmement, vous contestez l'extension de l'usage des scanners à ondes millimétriques, y compris dans des lieux qui seraient sans lien avec les jeux Olympiques et Paralympiques. En réalité, l'article 11 du projet de loi s'inspire des dispositions applicables aux aéroports. Le recours aux scanners corporels est une mesure intrusive, il est vrai. C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit, bien évidemment, des garanties qui répondent aux exigences européennes

d'avoir accès à un autre dispositif de contrôle ; l'impossibilité pour l'agent d'identifier la personne contrôlée, puisque les images produites par les scanners correspondent à des représentations banalisées du corps humain ; le brouillage de la visualisation visualisation du visage ; enfin, l'interdiction du stockage ou de l'enregistrement des images. Autant de garanties grâce auxquelles nous nous assurons que toutes les précautions seront prises afin d'éviter les dérives alarmantes que vous craignez tout autant que nous. Je précise également que cet article 11 permettrait de mettre un terme à une situation juridiquement alarmante, puisque d'autres portiques de ce type ont pu être installés par le passé sans faire l'objet de dispositions législatives autorisant ou encadrant leur usage. Quatrièmement, vous regrettez le recours toujours plus largement autorisé à une publicité visuelle envahissante, qui dénature selon vous les lieux comme les valeurs de l'olympisme. Certes, on peut regretter l'omniprésence quotidienne de la publicité sur les écrans. Mais considérer qu'autoriser un peu plus de publicité, pendant une période limitée, pour un événement tel que les Jeux, un événement tel que les Jeux, ce serait dénaturer les valeurs de l'olympisme, mes chers collègues, je crois que c'est un tantinet radical. Je rappelle que seuls les partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte, pourront bénéficier des nouvelles dérogations. Cela permettra notamment de limiter le financement public des Jeux en attirant et en conservant des partenaires privés, dans un contexte où la France souhaite organiser des Jeux raisonnables, y compris d'un point de vue financier. Cinquièmement, vous condamnez les dérogations au repos dominical dans une zone élargie qui serait sans justification ni lien avec la nature de l'événement sportif. Une fois encore, vos craintes sont injustifiées. En effet, la mise en oeuvre de la dérogation dérogation au repos dominical sera conditionnée au respect du volontariat des salariés, ainsi qu'à l'octroi des contreparties légales inscrites dans le code du travail. De plus, si les communes situées à proximité des sites de compétition ont été intégrées, c'est afin d'éviter un risque de rupture d'égalité entre les entreprises pour les communes qui, sans être limitrophes, auraient pu Enfin, vous justifiez le dépôt de votre motion par l'absence de questionnement ou de mesures portant sur l'héritage des Jeux, sur la manière dont les équipements sportifs seront rendus accessibles à la population et sur celle dont les Jeux pourraient redynamiser redynamiser nos politiques sportives. Mon cher collègue, je vous informe qu'un plan Héritage et Durabilité des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a été présenté en juin 2022. Je vous invite à le lire, car il témoigne du travail mené, qui est considérable et inédit en la matière. Ce travail se poursuivra afin de donner corps à des ambitions clairement définies en matière environnementale et sociale. Tony Estanguet le dit très bien Le nouveau modèle que nous construisons ensemble, ce sont des Jeux qui maîtrisent leur impact sur le territoire et sur la planète, des Jeux inclusifs et fédérateurs, des Jeux sobres et durables. En conclusion, mes chers collègues, j'espère vous avoir convaincus que la copie du Gouvernement n'a rien de néolibéral ou de techno-sécuritaire. Les mesures du projet de loi sont justifiées et proportionnées compte tenu de l'ampleur de l'événement. Parce que sécurité et liberté ne doivent pas être opposées et parce que les valeurs de l'olympisme doivent être préservées, je voterai contre cette motion et je vous invite, mes chers collègues, à en faire de même.

ce texte est attendu et nécessaire. Il comporte des mesures qui doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible pour que nous soyons au rendez-vous des jeux Olympiques et

mes chers collègues, parmi les vingt articles de ce projet de loi, trois enjeux se détachent particulièrement : la santé, la lutte contre le dopage et, surtout, la sécurité.

Pour rappel, jusqu'à 45 000 membres des forces de l'ordre pourraient être mobilisés. Notre responsabilité est de leur donner tous les moyens pour lutter efficacement contre la menace terroriste dans le respect des libertés publiques. Les articles 6 à 13 du projet de loi déploient les outils nécessaires sur ce sujet qui, à l'évidence, nécessite des moyens exceptionnels. En particulier, l'article 7 prévoit une innovation majeure pour le dispositif du maintien de l'ordre assisté par intelligence artificielle : il introduit dans le droit la possibilité d'avoir recours de manière expérimentale à ce que l'on qualifie de vidéosurveillance « intelligente » ou « augmentée », dispositif utilisant des algorithmes qui n'ont rien d'opaque afin d'identifier des situations potentiellement dangereuses, comme des mouvements de foule, l'objectif étant de gagner de précieuses minutes pour intervenir avant qu'un drame se produise. Je tiens à affirmer tout le soutien de mon groupe à ce nouveau moyen mis à disposition de nos forces de sécurité, qui a obtenu l'aval de la Cnil et du Conseil d'État. Je veux ici saluer le ministère de l'intérieur et ses services, mais surtout le remarquable travail de notre rapporteur Agnès Canayer, qui a su renforcer les garanties apportées pour atteindre le bon équilibre, en précisant

de juillet 2024, quelque 240 individus condamnés pour des faits de terrorisme seront sortis des prisons françaises. De l'aveu même du procureur national antiterroriste,

à Nice et à Londres afin d'évaluer les innovations réalisées avant les Jeux de Londres et de définir les conditions dans lesquelles nous pourrions développer, à titre exceptionnel, un système utilisant la reconnaissance biométrique en temps réel et garantissant une protection maximale tout en écartant, bien évidemment, tout risque de développement d'une société de la surveillance à la chinoise.

en matière de reconnaissance faciale, de définir collectivement un cadre comprenant des lignes rouges pour écarter tout risque d'atteintes aux libertés publiques, une méthodologie claire, par la voie expérimentale, et un régime exigeant et indépendant de contrôle renforçant singulièrement les pouvoirs de la Cnil. Bien évidemment, nous rejetons en bloc l'idée selon laquelle l'État pourrait avoir recours de manière usuelle à ce dispositif ou pourrait le pérenniser pour contrôler la population. Notre idéal français de liberté et d'égalité

permettant, par exception et de manière strictement subsidiaire, le recours ciblé et limité dans le temps à des systèmes de reconnaissance biométrique sur la voie publique, en temps réel, sur la base d'une menace préalablement identifiée

dont nous proposons qu'elle soit la Cnil, le nombre de caméras serait proportionné et l'on prévoirait la minimisation des données utilisées et leur sécurisation, une supervision humaine systématique, une traçabilité des usages et bien d'autres garanties que je ne développerai pas ici. En effet, ce n'est pas au détour d'un simple amendement sur ce projet de loi, dont l'écriture doit être techniquement affûtée pour rester dans le cadre constitutionnel et respecter les prescriptions de la Cnil et des instances européennes, que nous pourrons avoir un débat serein et argumenté. Je l'avais dit au ministre de l'intérieur Gérald Darmanin : ce débat aurait plutôt dû se tenir dans le cadre de l'élaboration

J'ai en mémoire l'attentat contre Charlie Hebdo. J'ai en mémoire l'intervention bouleversée et bouleversante de Dominique Estrosi Sassone après l'attentat sur la promenade des Anglais.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous entrons aujourd'hui dans la dernière ligne droite. Selon Montesquieu, « les desseins qui ont besoin de beaucoup de temps pour être exécutés ne réussissent presque jamais

Ce projet de loi procède à de nombreux ajustements visant notamment à accorder notre droit national au contrat conclu avec le CIO pour accueillir les Jeux en France. Nous attendons collectivement cette échéance avec impatience. Ce texte contient tout d'abord des mesures concrètes et novatrices en matière de lutte contre le dopage. On ne peut que s'en féliciter. Malheureusement, les auteurs de pratiques dopantes ont bien souvent une longueur d'avance sur le législateur. Ce texte autorise notamment les tests génétiques. La période qui suivra la fin des Jeux permettra de tirer tous les enseignements de cette pratique nouvelle. Je salue tout particulièrement l'ajout en commission de dispositions visant à rendre obligatoire la vente de billets d'accès infalsifiables pour les épreuves. Il s'agit précisément l'une des propositions phares du rapport des présidents de la commission de la culture et de la commission des lois dévoilé en juillet 2022. Les débordements que l'on a déplorés à la marge de la récente manifestation sportive organisée au Stade de France nous ont démontré toute la pertinence de cette mesure. Madame la ministre, cet ajout permettra- nous l'espérons -de sécuriser l'accès aux Jeux et aux zones de billetterie. Je souhaite également m'attarder sur les jeux Paralympiques. Ces épreuves vont bien au-delà du sport et de la performance individuelle, tant elles véhiculent des valeurs essentielles d'inclusion et de partage. La pratique du handisport ouvre aux autres, donne confiance en soi et permet aussi de retrouver une certaine autonomie. Nous devons veiller collectivement à donner à ces jeux Paralympiques la plus grande visibilité possible et à célébrer fièrement les quelque 4 400 athlètes qui concourront à partir du 28 août 2024. Je salue à ce titre l'implication sans failles de la Fédération française handisport, des clubs et des associations sportives. Les jeux Olympiques représentent aussi un formidable défi sécuritaire. Les grands rassemblements de personnes sont particulièrement menacés par le terrorisme, et nos services de sécurité sont mobilisés pour faire face à cette menace. Nous nous félicitons que ce projet de loi renforce leur efficacité, notamment avec la généralisation du criblage, qui resserre les mailles du filet et assure une plus grande sécurité à nos concitoyens. Il existe, en outre, des risques inhérents à ces grands rassemblements de personnes. Les mouvements de foule peuvent se révéler particulièrement dangereux. Pour prévenir ces risques, le projet de loi autorise la mise en oeuvre de technologies novatrices, afin de détecter les signes avant-coureurs de telles catastrophes. Nous saluons aussi la grande implication de la Cnil dans le développement de ces outils, ce qui augmente encore les garanties apportées par ce texte en matière de données à caractère personnel.

offrir une vaste célébration des valeurs du sport à nos concitoyens et aux 4 milliards de personnes qui suivront avec passion les Jeux aux quatre coins du globe. Je m'en remets désormais à la célèbre devise olympique, qui a déjà été citée, mais partiellement :, c'est-à-dire : :, c'est-à-dire : « plus vite, plus haut, plus fort -ensemble ». Espérons qu'elle guide les athlètes de l'équipe de France dans ces derniers mois d'intense préparation physique et mentale. La parole

est d'adapter notre arsenal juridique, du code du sport au code de la sécurité intérieure, afin de garantir une organisation fluide et sereine des jeux Olympiques de l'an prochain. Cependant, ce projet de loi va bien au-delà.

dans sa version initiale créent de nouvelles dispositions ou modifient des dispositions existantes de façon durable : pour une loi officiellement dédiée à un événement temporaire, cela peut nous alerter.

Jeux. Le déploiement de la vision sécuritaire et le recours massif, presque indifférencié, à la vidéosurveillance, le tout augmenté de mécanismes algorithmiques dangereux et potentiellement mis à disposition d'autres opérateurs ultérieurement, y compris non nationaux, soulèvent de nombreuses questions.

Se pose aussi la question du report de charge sur de nombreuses polices municipales : les fan zones des villes hôtes autres que Paris seront-elles sécurisées par la police nationale ? Pour les festivals et le monde de la culture, la dépense supplémentaire est particulièrement importante.

de la modification injustifiée des règles d'ouverture dominicale : sous prétexte d'une temporalité courte et de la volonté de bénéficier d'un pic de consommation, le Gouvernement ouvre la porte à de nouvelles dérogations au droit du travail. Le recours au bénévolat est, lui aussi, très problématique, tout autant que le recours au secteur privé ou la concentration des moyens des forces de sécurité nationale, qui posent également la question du respect du droit du travail. La Cour des comptes estime qu'il faudrait employer 22 000 à 33 000 agents de sécurité privée par jour pour sécuriser l'ensemble des épreuves. Ces chiffres dépassent largement les capacités disponibles dans les entreprises de la région et du pays. La question de la formation et du recrutement de ces agents n'a pas été anticipée. Le spectre de l'expérience londonienne et de l'explosion des coûts n'est pas si éloigné.

L'héritage de ces Jeux, au centre des préoccupations affichées du comité d'organisation, n'est pas davantage environnemental, malgré les annonces et les efforts locaux. À Marseille, par exemple, sans le travail de la ville, l'ambition et les actions pour la préservation et la reconstitution de l'écosystème marin en bord de mer n'auraient pas été les mêmes. Ce texte est les mêmes. Ce texte est à l'image des tentatives de ces dernières années d'ériger la surveillance de masse en clé de sécurité et de justifier les renoncements aux libertés individuelles et collectives par des arguments sécuritaires. Cette vision, surtout lorsqu'elle tente de s'habiller des habits consensuels du bon déroulement des jeux Olympiques,

des citoyens. Aussi, faute de modifications significatives, particulièrement sur la temporalité de l'application des mesures qui y figurent, notre groupe votera contre ce projet de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans quelques mois, la France accueillera, pour la première fois depuis près d'un siècle, les jeux Olympiques et Paralympiques d'été. Du 24 juillet au 8 septembre prochains, 14 850 athlètes, répartis en 388 délégations et 58 sports, s'affronteront dans le cadre de 878 épreuves. Plus de 11 millions de spectateurs, venus du monde entier, sont attendus sur les différents sites de la compétition et à leurs abords. Ils seront 4 milliards derrière leur écran. C'est une compétition populaire aux enjeux inédits. La France doit être au rendez-vous de ces Jeux ; c'est là tout l'objectif de ce texte. Le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 doit ainsi permettre à notre pays de répondre de la manière la plus adéquate possible aux défis que pose l'organisation d'un tel événement. Il vise ainsi à satisfaire de nombreux besoins en matière de sécurité, de couverture sanitaire, de lutte contre le dopage, de formation aux gestes qui sauvent ou encore de mobilité inclusive.

Il doit être examiné au regard de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, que nous avons adoptée le 14 décembre dernier, et qui prévoit des moyens exceptionnels en matière de sécurité des différents sites. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui parachève ce cadre législatif. Les sources de satisfactions y sont nombreuses. Ainsi, la mise en oeuvre de certaines mesures, à commencer par l'ouverture le dimanche des commerces situés à proximité des sites de compétition, devrait permettre aux acteurs économiques de profiter de retombées considérables et constituer un véritable accélérateur d'investissement. D'autres contribueront à limiter le financement public. Ce sera notamment le cas, à l'article 14, de l'extension de la dérogation légale aux interdictions de publicité dans l'espace public. Nous constatons également avec satisfaction que les dispositifs dérogatoires et expérimentaux ont été assortis de nombreuses garanties. Nous nous réjouissons en particulier que la ligne rouge de la reconnaissance faciale n'ait pas été franchie. Ce projet de loi nous donne par ailleurs l'occasion de mettre notre droit en conformité avec le code mondial antidopage et le droit européen sur la protection des données. Je pense notamment aux tests génétiques aux fins de lutte contre le dopage, à l'article 4, et au cadre légal de la vidéoprotection, à l'article 6. Autre motif de satisfaction, certaines dispositions contenues dans ce texte ont un caractère permanent. permanent. Je pense ainsi à l'introduction de deux nouveaux délits dans le code du sport, ce qui permettra de lutter plus efficacement contre les infractions commises lors de compétitions sportives. Nous nous félicitons enfin de constater que certaines mesures entreront en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi au. Le laboratoire Le laboratoire antidopage français, la SNCF, la RATP et les organisateurs disposeront ainsi du temps nécessaire pour tester et adapter les nouveaux dispositifs que sont les analyses génétiques, les caméras augmentées ou l'application de la procédure de criblage aux fan zones et aux participants aux grands événements. La commission des lois a adopté une trentaine d'amendements, qui sont de nature à consolider ce texte. Le renforcement des garanties entourant l'expérimentation des traitements algorithmiques d'analyse automatisée des images de vidéosurveillance est ainsi bienvenu. Il va dans le sens des recommandations formulées par le Conseil d'État et la Cnil. En ce qui concerne l'encadrement des tests génétiques aux fins de lutte contre le dopage, la rapporteure Canayer propose d'inscrire l'ensemble du dispositif dans le code du sport. Nous n'y voyons

à la lutte contre le dopage. Mes chers collègues, ce projet de loi est un texte nécessaire ; nous avons aussi souhaité en faire un texte équilibré. Je vous invite à l'adopter pour faire des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 une réussite française, un succès pour le monde sportif et pour nos athlètes,

Candidature déposée sous la présidence de François Hollande, victoire décrochée sous la présidence d'Emmanuel Macron : cet événement dépasse les clivages. À droite comme à gauche, on a considéré qu'il ne fallait pas politiser les candidatures visant à accueillir les événements sportifs- si vous me permettez de paraphraser Emmanuel Macron Nous sommes donc spontanément favorables à ce texte, car nous souhaitons la réussite des jeux Olympiques et Paralympiques. Le groupe socialiste n'a d'ailleurs pas jugé bon de déposer des amendements sur un certain nombre de dispositions, qui ne posent pas problème. quelques sujets d'inquiétude demeurent. Ainsi, nombre d'articles de ce texte prévoient des mesures destinées à s'inscrire de manière pérenne dans le droit commun ; d'autres visent à mettre en place des expérimentations et d'autres encore concernent bien exclusivement les jeux Olympiques et Paralympiques. Cela nous incite à nous interroger sur l'application de l'article 45 de la Constitution : en pareil cas, il nous semble bien délicat de définir précisément le périmètre du texte. À cet égard, je remercie la commission des lois de nous avoir octroyé une victoire symbolique en rebaptisant ce texte comme portant « diverses autres dispositions ». Je regrette cependant que ne figurent, parmi ces diverses autres dispositions, ni le montant de la taxe de séjour pendant les jeux Olympiques ni la privatisation du réseau de bus parisien. La situation catastrophique des transports en commun franciliens peut perdurer jusqu'en 2024. La privatisation va-t-elle empirer les choses ? « Je ne vous ferai pas croire que nous n'y pensons pas reprendre les termes du ministre des transports, Clément Beaune. Hélas, nous ne pourrons nous prononcer sur cette situation dans cet hémicycle, puisque les amendements du groupe socialiste sur ce sujet, qui a pourtant tout à voir avec l'objet de ce projet de loi, ont été déclarés irrecevables. Ensuite, ce projet de loi, qui ne parle pas que des Jeux, tout en en parlant, mais sans ne parler que de cela, autorise nombre d'expérimentations. Notre premier souci que des garanties suffisantes soient apportées pour maîtriser les dérogations dans leur périmètre, dans leur durée et dans leur objet, et qu'elles soient ainsi parfaitement cadrées. Le Conseil d'État avait proposé au Gouvernement un vade-mecum de l'expérimentation tant il est rare qu'une expérimentation ne soit pas généralisée. Est-ce à dire qu'elles sont toutes extrêmement efficaces et convaincantes ? Il est permis d'en douter ... Le Conseil d'État a donc recommandé au Gouvernement de définir, en amont des expérimentations, des critères de réussite et des objectifs clairs tout en associant le plus largement possible le public concerné. Après avoir lu l'étude d'impact de ce projet de loi, nous doutons de la définition de ces quelques critères. Mme la ministre serait-elle, par exemple, en capacité de me dire ce qui pourrait conclure à la non-généralisation de l'utilisation de la vidéoprotection automatisée ?

Il est bien difficile de leur rétorquer qu'ils se trompent et que les mesures proposées ne sont que temporaires. À travers les auditions de la commission, nous avons eu la confirmation que beaucoup d'acteurs se projettent déjà dans une pérennisation. Je ne dis pas que cela est incompréhensible, mais ne serait-il pas plus transparent d'indiquer, dès le départ, que la plupart des mesures proposées sont en réalité destinées à durer ? C'est aussi l'une des raisons qui nous ont poussés à rejeter la reconnaissance faciale. Nous considérons que le sujet n'est pas anodin et qu'il mérite un débat et une expérimentation assortie de garanties élevées d'encadrement pour rendre le dispositif acceptable. On ne peut introduire dans le droit positif des dispositions aussi lourdes par le biais d'amendements à un texte qui concerne les jeux Olympiques et Paralympiques. L'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale sont déjà présentes dans nos vies, la plupart de nos concitoyens en sont conscients. Faut-il donc leur faire croire que ce sont les Jeux de Paris qui rendent l'expérimentation technologique nécessaire ? Nous devons veiller à ce que le combat contre le terrorisme, bien légitime, ne conduise pas à des restrictions de libertés en matière d'ordre public. Il convient aussi de ne pas favoriser l'extension

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ces jeux Olympiques auraient pu, auraient dû donner lieu à un élan exceptionnel en faveur d'une politique sportive ambitieuse et populaire. visant à démocratiser le sport en France n'y a malheureusement pas répondu et ce nouveau texte n'apportera rien en la matière. Pis, celui-ci semble servir de soupape au Gouvernement pour prendre un certain nombre de dispositions restreignant les libertés individuelles et collectives appelées à s'appliquer de façon pérenne. Ce projet de loi aurait pu être l'occasion d'un débat positif sur la méthode à adopter pour que la prochaine Coupe du monde de rugby ou les jeux Olympiques de Paris constituent un héritage économique et social vertueux pour la population. Au-delà de la performance de nos athlètes et de la bonne tenue de l'événement en matière de sécurité et de transport, ces Jeux ne seront une réussite que s'ils permettent de casser les barrières sociales, territoriales et liées aux handicaps entre les usagers et la pratique sportive. Et comment concevoir un héritage économique pour nos collectivités en matière d'équipements alors même qu'elles peinent à soutenir leur vie associative ou à maintenir ouverts leurs équipements existants du fait de la hausse des coûts de l'énergie ? Que l'on se comprenne bien : je suis résolument pour la tenue de ces jeux Olympiques dans notre pays. La promotion faite au sport d'élite ne me gêne pas et les bonnes performances de nos athlètes nous honoreront. Ainsi, à défaut d'un héritage social, nous devrons nous satisfaire d'un héritage sécuritaire des Jeux. Loin de nous l'idée de négliger la sécurité de millions de femmes et d'hommes venus assister aux festivités, mais les dérogations apportées au droit commun en matière de droit des justiciables risquent de saper l'élan populaire que doit amener cet événement mondial. L'un des objectifs de ce texte est de légaliser la vidéosurveillance algorithmique. Or celle-ci a tout autant recours que la reconnaissance faciale à l'analyse biométrique, autrement dit à la détection de corps pour repérer ou identifier une personne. Étape par étape, la population est préparée à devoir accepter ces nouvelles technologies, sous couvert de leur caractère exceptionnel et limité dans le temps, alors même que ce gouvernement a la fâcheuse tendance d'inscrire de manière pérenne dans le droit commun

plus près. Ce texte de loi, en sus de n'apporter aucune garantie supplémentaire de bonne gestion de l'événement pour les supporters dans les stades, s'inscrit dans une ligne du tout sécuritaire qui nous semble contre-productive. Nos amendements tendent à corriger cette orientation, notamment en matière de pointage. En effet, nous estimons nécessaire de proportionner cette mesure au regard du comportement de la personne. personne. S'agissant de la pyrotechnie, les supporters, partout dans le monde, utilisent des torches et des fumigènes pour animer les tribunes. Bien qu'elle soit interdite, cette pratique perdure. Or la répression a des effets opposés à ceux

Faute d'une préparation sérieuse, nous en sommes amenés à devoir faire appel aux réserves de la police, de la gendarmerie et des armées. Entre les festivals de musique annulés, faute d'agents de sécurité publique et de membres des forces armées assurant le maintien de l'ordre public, je peine à distinguer l'horizon d'une quelconque communion populaire lors de ces Jeux.

il renforce la sécurité des Jeux et des grands événements que la France accueille. Le chapitre III, au gré des mesures importantes de sécurité qu'il implique et du traitement des questions, parfois épineuses, qu'il soulève, mérite une attention particulière,

Quelques imprécisions ou imperfections ont été relevées dans le texte du projet de loi, notamment le fait que l'installation de systèmes de vidéoprotection n'aurait été réalisable que « dans les moyens de transport et les voies les desservant ». Je me félicite

de vidéoprotection. Il est vrai que ces rapports ne sont plus rendus à la Cnil depuis 2013, ce qui emporte assez peu de conséquences pratiques.

Même quand cela n'arrange pas, la règle doit être respectée. Il est possible d'anticiper des nominations, il est possible d'anticiper des limites d'âge, il pourrait même être organisé des tuilages avec des adjoints ... Excellent ! C'est pourquoi nous exprimerons notre hostilité à un amendement d'Ancien Régime, très « versaillais

je salue, madame la ministre, le fait que vous ayez suivi l'avis du Conseil d'État. En effet, celui-ci suggérait, au nom de l'égalité entre les entreprises, d'étendre le périmètre géographique de la mesure aux communes situées à proximité des sites de compétition et non de le restreindre aux seules communes d'implantation de ces sites et aux communes limitrophes. Nous saluons, d'une manière générale, le travail de la rapporteure Agnès Canayer, qui a permis de trouver un équilibre. Je pense notamment à l'article 4 relatif à la lutte contre le dopage qui prévoit la réalisation d'analyses par des examens génétiques. La solution trouvée, permettre une expérimentation des tests génétiques les plus intrusifs, me paraît plus raisonnable sur le plan éthique. De même, nous souscrivons aux garanties apportées par la commission des lois à l'installation de scanners corporels à ondes millimétriques, basées sur le volontariat à la fois des gestionnaires et des personnes contrôlées, auxquels on ne pourra imposer ce dispositif. Nous doutons cependant de la portée pratique de cette faculté au regard de la capacité des opérateurs à investir dans ces machines coûteuses et à disposer d'agents formés. Enfin, Enfin, si nous reconnaissons l'utilité de ce projet de loi, nous aurions aimé qu'il ne subisse pas, lui aussi, la sentence d'une procédure accélérée qui nuit au temps du dialogue et du débat nécessaires au bon fonctionnement démocratique. démocratique. C'est aussi parce que ce texte ne peut, faute de temps, faire l'objet de discussions plus approfondies, que nous saluons la décision du Gouvernement et celle de la commission des lois de ne recourir à l'intelligence artificielle qu'à titre expérimental et de manière limitée, dans le temps et dans l'espace, le tout dans un cadre très contraint et sans aucune utilisation de données biométriques.

et me réjouir de la tenue des jeux Olympiques sur notre territoire. J'aurais aimé faire comme si tout allait bien, comme si l'on pouvait circuler normalement en Île-de-France, comme si les transports en commun étaient fonctionnels et sans danger. La vérité est que je peine à imaginer Paris en pleins Jeux, alors que nous avons déjà tant de mal à sécuriser un match de football. Rappelez-vous, madame la ministre, l'épisode du fiasco du Stade de France le 28 mai dernier. On peut espérer que le nouveau préfet évitera le pire et assurera mieux la sécurité des 13,5 millions de spectateurs attendus.

L'article 7 prévoit le recours aux caméras augmentées utilisant l'intelligence artificielle, ou vidéosurveillance algorithmique (VSA), afin de détecter des « situations anormales ». On parle alors d'une technologie qui analysera, classera, évaluera nos moindres faits et gestes dans l'espace public. La Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur internet, dénonce « une véritable frénésie sécuritaire » et « un projet totalement dystopique le Conseil d'État juge que le projet de loi est « susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d'autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d'aller et venir et les libertés d'opinion et de manifestation, lorsque ces dernières s'exercent à l'occasion de ces événements ». Il appelle l'intervention du législateur pour encadrer le texte de garanties rigoureuses. Et ce d'autant plus que nombre des mesures concernant la sécurité ont vocation à se pérenniser dans notre droit commun, dépassant ainsi le strict cadre des jeux Olympiques. nous montrer particulièrement attentifs et trouver le juste équilibre entre sécurité et protection de nos libertés. N'oublions pas non plus

Il faut tout faire pour que le sport sorte vainqueur de cette compétition, bien au-delà de la seule réussite commerciale de cet événement planétaire.

Notre pays doit être à la hauteur de ces jeux Olympiques et Paralympiques par la maîtrise des coûts de l'organisation, par la sécurité due aux athlètes et aux spectateurs et, enfin, par l'héritage que doit léguer cet événement.

Le coût réel des Jeux comprendra aussi les dépenses des collectivités territoriales et les dépenses de l'État relatives au dispositif de sécurité autour de l'événement et au sein des infrastructures de transport.

Madame la ministre, vous avez fait part de vos objectifs : vous voulez que les jeux laissent « une empreinte durable, tout d'abord matérielle, notamment en Seine-Saint-Denis, avec la construction d'équipements sportifs de proximité, de 4 000 logements accessibles ou d'aménagements routiers, piétons ou vélos d'utilité publique Nous veillerons à la réalisation de ces objectifs, auxquels nous adhérons. En ce sens, la commission de la culture a adopté l'amendement de son président Laurent Lafon visant à mutualiser les moyens de la Solideo avec un autre établissement de l'État. Cela devrait permettre à la société de se maintenir durant la phase de reconversion des ouvrages en s'appuyant sur les moyens d'un autre établissement public foncier et d'aménagement.

des forces de l'ordre seront mobilisés chaque jour pendant les épreuves et leur présence dans les transports en commun sera doublée. Nous regrettons que l'amendement de notre collègue du groupe RDSE Nathalie Delattre n'ait pas été retenu. Il visait à s'assurer que les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité- nous approuvons cette démarche -retrouvent, après l'événement, leur affectation antérieure au plus tard le 31 décembre 2024. En effet, durant la période des Jeux, aucune compagnie de CRS maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) ne sera affectée sur les plages, du fait de leur mobilisation sur les sites olympiques. De nombreux élus craignent les conséquences de cette absence, associée à un afflux majeur de touristes. Ils redoutent aussi que l'absence des compagnies de sécurité sur les plages ne devienne pérenne. J'en viens à l'héritage immatériel que devront laisser les jeux Olympiques et paralympiques de 2024. Au-delà du rayonnement touristique de la France, ils sont une formidable opportunité pour promouvoir la pratique sportive, par la mise en lumière non seulement de disciplines encore confidentielles dans d'autres pays, du handisport et du sport féminin, dont nous célébrons aujourd'hui même la journée internationale. Plus généralement, les Jeux sont un encouragement à la pratique sportive pour tous, une source d'épanouissement, d'apprentissage et de respect des règles, des arbitres et des adversaires, autant de valeurs que notre pays a bien besoin de rappeler.

Loin de l'élitisme social de ses origines et du « sport business » actuel avec ses « athlètes produits », il puise dans l'esprit olympique un équilibre entre la promotion de l'activité physique et les valeurs de respect et de fraternité. Enfin, je salue la décision de conserver France Télévisions comme diffuseur officiel des jeux Olympiques. À l'heure où certaines rencontres sportives disparaissent des chaînes du service public, il est bon

les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ne se limitent pas à la seule capitale. Plusieurs autres villes se sont engagées à accueillir des compétitions, des centres de préparation, les villages des athlètes et des médias ou encore le parcours de la flamme.

Or, à dix-huit mois du début des compétitions, force est de constater que l'enthousiasme de la population française reste pour le moins mesuré, les Français devant, pour l'heure, faire face aux crises sanitaire, sociale et de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il est donc de notre responsabilité collective- Cojop, État, Parlement, collectivités, grande famille du sport français -de tout faire pour préparer dans les meilleures conditions l'organisation et l'accueil de la plus grande compétition sportive planétaire.

des délais serrés pour la livraison de toutes les infrastructures, une organisation loin d'être dans les clous concernant l'offre de transport qui ne pourra, à ce rythme, être prête à temps, et des questions de sécurité évidentes auxquelles ce projet de loi est, à raison, largement consacré.

des mesures antidopage qui, une fois pérennisées, constitueront un héritage durable de ces Jeux. Nous pouvons en être fiers. Il y avait en effet urgence à adapter des dispositifs complémentaires en matière de gestion des grands événements. Vidéoprotection, contrôle des entrées, renforcement des sanctions pour les faits de violence ou de fraude, sécurité dans les transports ... le texte se veut tout terrain. Encore faut-il bien délimiter le périmètre des mesures exceptionnelles et celui des changements permanents. Aussi, nous sommes favorables à ce texte qui, je l'espère, nous permettra d'éviter un nouveau fiasco semblable à celui du Stade de France, devenu le symbole de tous les dysfonctionnements possibles lors d'une rencontre internationale.

L'absence de garanties sur leur accueil, qui révèle des enjeux propres à l'événement- logements peu accessibles en Île-de-France et dans Paris intra-muros -, ou l'absence de facilités de transport peuvent créer un sentiment d'exclusion, à l'opposé des valeurs de l'olympisme. Faut-il rappeler que, au-delà des chiffres, des femmes et des hommes consacreront leur temps et leur énergie à faire de ces Jeux une réussite à tous les niveaux ? Ils doivent pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Le dispositif des volontaires, les conditions de candidature, les rôles assignés à chacun sont inscrits dans la charte du volontariat olympique et paralympique que nous devons à la loi de 2018. Pour la grande majorité des bénévoles, il s'agit d'un cadre sain, clair, qui les protège autant qu'il protège les spectateurs. Mais, là encore, des doutes persistent : quelle est la valeur contraignante d'une charte pour des profils dangereux qui souhaiteraient à tout prix gâcher la fête ? ? En l'état, ni l'organisateur ni le Gouvernement n'apportent de réponse satisfaisante. Par ailleurs, le Premier président de la Cour des comptes appelle à une nécessaire vigilance face aux risques juridiques associés à la charte du volontariat olympique,

y tient : les billets seront nominatifs. Or les partenaires comme la Ville de Paris, la région Île-de-France, les entreprises et les associations, la billetterie sociale, se feront les acquéreurs de places pour inviter du public. À quel nom seront ces billets ? Comment s'assurer que les personnes se présentant avec un billet en sont bien les propriétaires ? Comment effectuer les contrôles ? Sans réponse précise à ces questions pourtant pratico-pratiques, tous nos grands débats seront vains. Le billet d'entrée n'est pas un objet ordinaire : il est la clef d'accès à l'expérience olympique pour des millions de personnes venues du monde entier. Pour beaucoup de jeunes, c'est aussi le sésame vers une première rencontre avec le sport de haut niveau. Madame la ministre, de ces jeux Olympiques et Paralympiques, l'important n'est pas uniquement de participer, mais de s'assurer de leur succès. Il faut agir « plus vite, plus haut, plus fort »- et j'ajouterai : ensemble !

La réussite des Jeux de 2024, événement tout à fait exceptionnel, est un enjeu majeur auquel nous adhérons collectivement. Pendant six semaines, 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs sont attendus. L'équivalent de cinquante-quatre championnats du monde seront organisés simultanément et circonscrits à un même lieu, ou presque. l'événement se mesurera à l'aune de son organisation, des résultats de nos athlètes, du respect de l'équilibre budgétaire- il s'agira de limiter les dépassements au maximum -, des retombées économiques et sociales, en termes d'infrastructures- la notion d'héritage olympique doit être hiérarchisée -, à l'aune également de ses dimensions festive, inclusive, populaire, environnementale, mais aussi du rayonnement de la France et de la valorisation de ses règles communes et de ses savoir-faire.

Présentées comme nécessaires, ces dérogations permettent en effet d'appliquer le cahier des charges du CIO, de respecter la Charte olympique, de mettre en oeuvre les contrats de ville hôte et d'harmoniser, dans notre législation, les standards de l'Agence mondiale antidopage- je fais ici référence aux tests génétiques déjà appliqués aux Jeux de Tokyo en 2021. Nous notons que le Gouvernement a globalement respecté l'essentiel des recommandations du Conseil d'État et de la Cnil. Parallèlement, le projet de loi regroupe un ensemble de dispositions pérennes ou amenées à l'être après expérimentation et/ou évaluation, et qui dépassent largement le cadre olympique, en s'appliquant potentiellement à « des manifestations récréatives, sportives et culturelles » ayant lieu avant et après 2024 Coupe du monde de rugby 2023, concerts, festivals ... Les décrets d'application définissant la nature des événements concernés ou les seuils retenus seront l'objet de notre particulière attention. C'est en ce point que réside la dimension post-olympique du texte, absente d'un intitulé réducteur, bien que précisé en commission. Concernant l'aspect sécuritaire, il semble que les enseignements des incidents survenus lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai dernier aient été globalement tirés par les ministères concernés, par la Cependant, deux situations sensibles sont identifiées : la cérémonie d'ouverture et le parcours de la flamme olympique dans le pays. La gestion de la cérémonie d'ouverture paraît d'une grande complexité et nécessite un haut degré d'anticipation, des moyens accrus et un niveau de technicité auquel nous n'avons jusqu'alors jamais recouru. Des arbitrages rapides sont nécessaires afin de susciter la sérénité dans l'opinion publique. Ces choix stratégiques intègrent également la gestion des risques d'atteintes aux personnes et aux biens, ainsi que la politique de la délinquance du quotidien aux abords des sites accueillant des compétitions, qui pourraient menacer le caractère paisible de l'événement.

des jeux Olympiques de Paris 2024 reposera en grande partie sur l'équilibre que nous parviendrons à trouver entre la quiétude que nous devons aux habitants, spectateurs et participants et le souci de préserver la dimension fédératrice et festive de l'événement. La discussion

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 1 crée la polyclinique olympique et paralympique prévue par le contrat de ville hôte. Nous avons bien compris que la création de cette polyclinique, sous forme de centre de santé, vise à préserver la bulle sécuritaire athlètes, le village olympique et paralympique, mais aussi à ne pas reporter des besoins propres à ces derniers sur l'offre de soins de la région. En pratique, la polyclinique sera gérée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et nous espérons vivement que les dépenses qu'elle engagera seront intégralement remboursées par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 2024. Le fonctionnement de ce centre devrait reposer sur un encadrement soignant assuré par des praticiens de l'AP-HP. Toutefois, l'essentiel des professionnels de santé qui y exerceront seront des volontaires olympiques et paralympiques. et paralympiques. Les besoins médicaux, paramédicaux et administratifs du pic d'activité sont estimés à 193 volontaires. Compte tenu de l'état de nos hôpitaux publics, à Paris comme ailleurs, il ne faudrait pas déshabiller Pierre pour habiller Paul

d'autant plus que trois hôpitaux participeront également à la prise en charge des soins outrepassant les compétences du centre de santé olympique. Beaucoup de questions restent en suspens. Plus globalement, la saturation des capacités d'accueil des hôpitaux à la suite des fermetures de lits d'hospitalisation et du sous-investissement de l'État suscite notre interrogation quant à la prise en charge médicale et hospitalière des sportifs, des journalistes et, bien évidemment, des supporters et touristes durant les prochains Nos hôpitaux publics sont en grande souffrance, peut-être encore davantage pendant les périodes estivales, à Paris comme ailleurs. Aussi aimerions-nous que le Gouvernement nous rassure sur tous ces points.

Les hospitalisations et les actes chirurgicaux seront en effet du ressort des hôpitaux Bichat, Avicenne et Pompidou. En outre, la dénomination « centre de santé » correspond au statut juridique de l'établissement de santé qui prendra en charge les patients du village olympique et paralympique. Quel

pas de tiers payant, puisque les actes seront réalisés à titre gratuit et financés par Paris 2024 ; l'exercice salarié n'y est pas promu non plus, puisque, outre l'encadrement salarié de l'AP-HP, les praticiens qui y exerceront seront des volontaires olympiques.

de l'ensemble des dépenses engagées pour ce centre de santé spécifique et de la prise en charge des athlètes et personnes accréditées qui seraient éventuellement orientées par ce biais au sein de l'AP-HP. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter cette phrase redondante

la ministre, la capacité du système de santé de la proche couronne parisienne à faire face à l'afflux de population et nécessairement à l'afflux de demande de soins Il faut que vous nous répondiez maintenant et que vous nous disiez quelle est la programmation de votre ministère pour satisfaire cette demande supplémentaire. Votre collègue, M. Darmanin, nous a dit de façon extrêmement claire et tout à fait honnête que les agents des forces de police n'auraient pas de vacances en juillet et en août 2024. Estimez-vous qu'il en sera de même pour les personnels de santé ?

sur les capacités de l'offre de soins francilienne à répondre aux besoins identifiés pour la période des Jeux de Paris 2024. Une demande de rapport ne me semblant ni opportune ni nécessaire, je suis défavorable

M. Jérémy Bacchi. L'article 17 du projet de loi prévoit que, dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le préfet peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de

Les conséquences du travail le dimanche sur la santé, la sociabilité, la famille, les relations amicales et les loisirs sont pourtant connues. Les compensations financières et en jours de repos ne suffisent pas aux travailleurs Par conséquent, nous refusons toute nouvelle dérogation au repos dominical, laquelle entraînerait nécessairement une dégradation de l'état de santé des travailleuses et des travailleurs, déjà profondément affectés. Quel La commission a considéré que la dérogation au repos dominical prévue à l'article 17 était justifiée par les besoins des visiteurs et des travailleurs présents pendant les Jeux et suffisamment encadrée dans le temps et dans l'espace. En outre, des garanties sont apportées aux salariés concernés. Nous sommes donc défavorables à la suppression de cet article.

car tous les départements ne sont pas concernés par les épreuves olympiques et paralympiques. La loi Macron de 2015 permet déjà de déroger au repos dominical dans les zones commerciales, dans les zones touristiques, dans les zones touristiques internationales et dans les gares. En outre, les maires ont la possibilité de fixer une liste de douze dimanches par an permettant aux commerces de détail de déroger au repos dominical-

selon les territoires, l'affluence du public pourra se trouver dans la commune d'implantation des sites de compétition, mais aussi dans des communes limitrophes ou situées à proximité en raison des infrastructures de transports, des capacités hôtelières ou encore des sites touristiques qui s'y trouvent. Laissons la possibilité aux préfets d'autoriser certains commerces à ouvrir le dimanche dans les communes limitrophes ou situées à proximité des lieux de compétition pour s'adapter au mieux aux besoins des visiteurs.

Ainsi, des autorisations collectives pourraient être délivrées pour plusieurs établissements afin, prétendument, de répondre aux besoins du public.

y sommes défavorables, puisque plusieurs communes étant susceptibles d'être concernées pour un ensemble d'établissements qui répondent aux besoins d'un même public, il apparaît plus pertinent de maintenir la compétence du préfet pour délivrer les autorisations. Je rappelle que la dérogation proposée ne se substituera pas

bienvenue : de nombreuses demandes seront à traiter, les besoins du public sont déjà largement prévisibles et la dérogation est bien encadrée. Il n'est pas souhaitable de revenir sur cette simplification. La commission est donc également

Cette nouvelle dérogation s'ajoute à celles qui existent déjà au titre des zones touristiques internationales, pour Paris au moins, des zones touristiques et des dimanches dits des maires. Du fait de ce dernier dispositif dérogatoire, la période des soldes d'été 2024, donc le mois de juillet, est déjà ouverte au travail le dimanche. En outre, si l'on retient la durée initialement prévue dans le projet de loi, ce sont

De nombreux visiteurs, touristes et travailleurs sont attendus avant, pendant et après les Jeux. Pour ces touristes français et étrangers qui vont venir visiter le pays et pour les travailleurs mobilisés en amont

avec beaucoup de bienveillance : nous sommes ensemble pour deux jours, nous sommes tous partisans des jeux Olympiques, mais vous devez nous aider

professionnelle et vie familiale, il convient, comme pour les dates modificatives des dimanches dits du maire, que l'autorisation intervienne au moins deux mois avant le premier dimanche susceptible d'être travaillé. Cela est d'autant plus important que cette

et l'application de la dérogation au repos dominical ne me semble pas nécessaire. Il est préférable que le Gouvernement précise par instruction, en lien avec les services des préfectures, les délais d'examen des demandes et la manière de les anticiper au mieux pour les employeurs et les salariés. Il pourra aussi être utile que le préfet puisse adapter les autorisations de dérogation en cas d'évolution des besoins du public, si la situation le nécessite. Il n'est pas souhaitable que la loi fixe tous les détails de la procédure.

Le préfet doit pouvoir suspendre à titre temporaire les arrêtés de fermeture hebdomadaire applicables dans certaines professions s'ils rendent impossible l'ouverture dominicale des commerces concernés.

Madame la ministre, d'apprécier au mieux les besoins locaux, avec l'avis de toutes les parties prenantes. Nous ne voulons pas contraindre à l'excès ce travail d'instruction et de concertation mené par les préfets. Pour ces

en application du code du travail, au cas par cas, selon les secteurs géographiques concernés, et avec toute la marge d'appréciation nécessaire pour tenir compte de la volonté exprimée par les organisations d'employeurs et de salariés.

Le projet de loi avait initialement prévu une expérimentation générale en matière de tests génétiques. La commission des lois avait opéré un premier distinguo entre les tests visant à réaliser une comparaison d'empreintes génétiques, qu'elle pérennise, et ceux qui permettent d'analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.

tout de même retenu la voie prudente de l'expérimentation, tout en introduisant deux modifications importantes, qui étendaient considérablement le périmètre et la durée d'application de l'article 4.

de l'expérimentation et le rapport d'évaluation pour en tirer les conclusions qui s'imposent. Quel

et de transmission des informations reçues en vue d'orienter les investigations antidopage. En amont, puis lors des Jeux, en sa qualité d'organisation nationale antidopage, l'AFLD est habilitée à mettre en oeuvre ces prérogatives pour établir et sanctionner les violations non analytiques des règles antidopage. Dans cette perspective,

informations à Tracfin, la réciproque n'a pas été prévue, ce qui nuit à l'efficacité des enquêtes antidopage en cours et à venir dans la perspective de 2024. C'est pourquoi cet amendement

Même si l'homologation est juridiquement nécessaire pour les peines de prison prévues par les lois du pays, il serait mal compris par les autorités polynésiennes

un certain nombre de clarifications importantes. La ministre de la culture a dit très clairement que, du 23 juin 2024

parallèlement aux jeux Olympiques et Paralympiques, durant l'été 2024, s'inscrivent dans la continuité de ceux de ma collègue Sylvie Robert. La présentation du dispositif des jeux Olympiques et Paralympiques au mois d'octobre dernier et l'annonce de l'obligation d'annulation ou de report de tous les événements nécessitant l'engagement d'unités de force mobile avaient suscité l'émoi des organisateurs de festivals et d'événements culturels. Je voudrais ici rappeler que le droit à la culture est un droit constitutionnel consacré par le préambule de 1946. Pour ces secteurs, qui peinent à retrouver leur public d'avant la crise, cette nouvelle incertitude est un coup dur. Dans le spectacle vivant, le pessimisme est toujours palpable, comme nous avons pu le constater à Nantes, le 13 janvier dernier, où se tenaient les biennales de la profession. La saison estivale offre des débouchés de diffusion indéniables à toute la filière- diffusion déjà fragilisée par l'attrition des budgets locaux du fait de la crise énergétique. L'instauration de nouvelles contraintes sécuritaires s'ajoute donc à une situation déjà critique. La circulaire du 13 décembre 2022 relative à la sécurisation des événements culturels, festifs et sportifs de l'été 2024 a le mérite de donner un cadre de programmation à tous les organisateurs, mais elle comporte en réalité plus de zones d'ombre que de réponses. Elle acte l'interdiction ou le report d'événements nécessitant la mobilisation d'unités de force mobile, qui seront toutes mobilisées pour la sécurisation des Jeux.

32 rectifié vise donc à réaffirmer que le maintien d'événements doit rester la règle et l'interdiction l'exception. C'est une formulation moins ambiguë que la « vocation à se maintenir » de la circulaire ... Il s'agit en outre d'inscrire ce principe dans la loi, plus stable juridiquement qu'une circulaire qui peut être facilement modifiée.

Il s'agit d'un critère difficile à appréhender à l'avance par les organisateurs : faut-il se fonder sur la sécurisation des événements passés ou sur l'état de la menace dans un an et demi pour des concertations et des programmations en cours ? Madame la ministre, pouvez-vous vous engager ici clairement à ce que tous les événements de moindre ampleur soient bien maintenus ? Il est également inscrit dans la circulaire que certains événements pourront bénéficier de dérogations, décidées dans le cadre national.

? Vous le voyez, la circulaire n'est pas claire ; et l'absence de clarté fragilise la liberté de création et le droit à la culture que j'évoquais précédemment. C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 33 tend à inscrire dans la loi des seuils qui puissent être opposables à chacun.

C'est un enjeu d'égalité territoriale. Il faut garantir une vie estivale locale riche à tous ceux qui n'auront pas la chance d'assister à des épreuves olympiques, éloignées de leur domicile. L'organisation d'événements culturels, festifs et sportifs est un levier indéniable d'attractivité touristique pendant la belle saison pour tous nos territoires. Il est donc absolument nécessaire

Là encore, si la circulaire du 13 décembre 2022 prévoit bien un dialogue avec les collectivités territoriales, le cadre n'en est pas clairement et juridiquement défini.

nous sommes très nombreux à nous inquiéter de la charge financière que représente l'organisation de ces jeux pour les collectivités territoriales.

Avons-nous collectivement conscience des implications d'un tel renversement ? Y souscrivons-nous ? Quelles garanties établissons-nous pour nous prémunir d'éventuelles fuites en avant ? Si l'argument utilitariste peut apparaître fondé au regard des menaces sécuritaires, il ne répond nullement à ces questions, qui concernent pourtant notre cadre commun d'existence. Si une telle solution technologique, qui complète un arsenal sécuritaire déjà fourni, limite le risque, elle ne l'efface pas. En d'autres termes, jusqu'où sommes prêts à rogner sur notre liberté pour préserver au maximum notre sécurité ? L'article 7 témoigne de cette recherche d'un équilibre particulièrement délicat à trouver. À cet égard, je salue le travail de la commission des lois

l'évaluation de l'expérimentation, compte tenu de son importance dans la perspective d'une éventuelle généralisation, doit présenter toutes les garanties d'indépendance qu'il est légitime d'attendre.

Nous devons muscler le continuum de sécurité pour enrayer les incivilités, la violence et l'insécurité qui règnent dans nos transports. C'était là tout le sens de nos amendements. Car on ne donne pas suffisamment de moyens aux acteurs de la sécurité dans les transports.

encore loin. J'espère que les prochains textes, notamment d'initiative parlementaire, permettront que la peur change enfin de camp

de surveillance globale. Les jeux Olympiques et Paralympiques ne sont ici qu'un prétexte pour jouer aux apprentis sorciers avec ces algorithmes de surveillance. Nous savons à quel point le marché est énorme.

nous a affirmé que l'objectif était d'éviter un « nouveau Séoul », en référence au drame ayant fait plus de 150 morts dans un mouvement de foule le soir d'Halloween, au mois d'octobre 2022. Mais sachez, chers collègues, que la Corée du Sud expérimente les caméras augmentées depuis

que vous évoquez. Le contrôle humain doit rester permanent pour nous assurer que ces algorithmes pourront détecter et signaler les événements prédéterminés et aideront nos forces de l'ordre à être plus efficaces et plus opérationnelles lors de l'organisation de grandes manifestations.

nous avons fait le choix d'accompagner le mouvement en déposant de très nombreux amendements. Si le premier travail d'encadrement qui a été produit par la rapporteure Agnès Canayer est déjà très sécurisant et solide, nos amendements visent à le renforcer ; la qualité de l'information du public ; la déclaration d'intérêt des prestataires extérieurs qui pourraient être appelés à développer ces systèmes ; le périmètre dans lequel ces systèmes pourraient être déployés ; l'effacement des données non pertinentes qui auraient été collectées pour ces systèmes

sur une durée limitée, ce qui pose un certain nombre de problèmes en termes de libertés publiques. Dans son avis du 8 décembre 2022, la Cnil estime que ces « outils d'analyse automatisée des images » peuvent « conduire à un traitement massif de données à caractère personnel ». Cela comporte

qui est révélateur des véritables intentions du Gouvernement : une fuite en avant techno-sécuritaire ! On veut gaver nos algorithmes de données. L'utilisation de ces dispositifs dans le simple cadre des jeux Olympiques et Paralympiques est, en soi, problématique. De tels délais

et nous en débattrons. Mais vous ne pouvez pas utiliser celui qui concerne les jeux Olympiques pour avancer toute votre machinerie sur la gestion algorithmique des populations.

de cette expérimentation, que d'aucuns ont d'ailleurs qualifiée de changement de paradigme, peut-être même civilisationnel. Je ne suis pas du tout convaincue

madame la ministre,

: La parole est à M. Bernard Fialaire. Le mécanisme que nous examinons ici n'a rien d'anodin, puisqu'il s'agit d'autoriser l'utilisation de traitements algorithmiques en matière de vidéosurveillance. Les bouleversements qu'introduit une telle expérimentation ont déjà été soulignés. D'ailleurs, la commission des lois en a conscience, puisque le texte qu'elle nous présente a déjà intégré des mécanismes de contrôle supplémentaires. Dans cette perspective, nous nous permettons de rappeler la prise de position de la Cnil, selon laquelle les « conditions d'application à cette nouvelle technologie des règles relatives à la protection des données et des principes protégeant les droits fondamentaux sont, en partie, incertaines ou à construire ». Aussi, face aux incertitudes, nous croyons que le dispositif doit être strictement limité et encadré. L'article 7 introduit deux conditions retenues alternativement, pour que le dispositif puisse être engagé : l'ampleur ou les circonstances de l'événement. Cependant, comme nous ne savons pas comment seront interprétés ces critères par les administrations et les juges, peut-être serait-il raisonnable dans un premier temps de les renforcer. Aussi proposons-nous d'ajouter une troisième le caractère exceptionnel de l'événement. Avec une telle condition, les rencontres hebdomadaires des compétitions nationales de football ou de rugby seraient exclues. En revanche, des matchs exceptionnels des matchs exceptionnels tels que la réception au Stade de France de la finale de la Ligue des champions au mois de mai dernier auraient pu entrer dans le dispositif.

l'usage. Pour y parvenir, nous proposons de rendre cumulatives les deux conditions d'ampleur et de circonstances qui permettent de désigner un événement. Nous le voyons bien, si ces conditions sont alternatives, les limites seront très difficiles à tracer ; on trouvera toujours une circonstance pour dire qu'il fallait activer le dispositif.

des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d'analyse dans l'espace public. La Cnil précise au passage qu'il est nécessaire d'empêcher tout phénomène d'accoutumance et de banalisation de ces technologies. Second problème, l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle est aujourd'hui dépourvue de cadre légal propre, dans le droit national comme dans le droit de l'Union européenne. Une proposition de règlement européen sur les systèmes d'intelligence artificielle est en cours d'élaboration, mais rien n'existe à l'heure actuelle. Ne nous leurrons pas devant l'objectif à peine voilé du Gouvernement d'étendre la portée de ces dispositifs par le droit : la durée extensive de l'expérimentation dont nous venons de débattre et le contenu du texte sont autant de preuves de la volonté de pérenniser ces expérimentations. Parce que nous refusons la banalisation de ces dispositifs sécuritaires, face au risque des dérives potentielles et dans l'attente d'une actualisation de la réglementation européenne, nous proposons d'inscrire expressément dans la loi que l'expérimentation n'a pas à être pérennisée d'office.

Même avis. Le Gouvernement a opté pour le principe de l'expérimentation, qui donnera lieu à une évaluation, donc à un passage, le cas échéant, devant le Parlement pour sa pérennisation.

le dispositif et d'avoir l'expérimentation la plus efficace possible.